La séance est reprise, la parole est à monsieur Bernard Jomier pour mise au point au sujet d'un vote. Merci monsieur le président, le groupe socialiste, écologiste et républicain souhaite procéder aux correctifs suivants concernant le scrutin public numéro 42 monsieur Jean-Claude Tissot souhaité voté pour cet amendement énonce abstenir je vous remercie. Acte est donné de votre mise au point, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés. Madame, monsieur le Ministre, mes chers collègues, la séance est reprise, nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 dans la discussion des articles que nous sommes parvenus à l'article trente-huit avec une prise de parole de Madame Cohen. Merci monsieur le Président, je voudrais profiter de l'article 38 pour intervenir sur la situation sanitaire à Mayotte que nous avons pu constater avec mes collègues de la commission des affaires sociales lors de notre déplacement en mars dernier, la situation économique, sociale et sanitaire de Mayotte est particulièrement difficile avec 34 % de la population qui renoncent aux soins pour un motif financier le seul hôpital de Mayotte à Mamoudzou est débordé et n'est pas en capacité de faire face aux besoins ni d'accueillir tous les patients dans des conditions satisfaisantes, le système de soins mahorais, bien qu'en expansion ne veut pas suivent la pression démographique, les soins se concentre ainsi de fait sur des activités non programmés les soins urgents : l'extension de la complémentaire santé solidaire à Mayotte est donc attendu pour mettre à niveau les droits sociaux et garantir le respect du droit fondamental à la protection de la santé, néanmoins je voudrais relayer les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment par l'association Médecins du Monde, qui alertent sur les ruptures de droits pour les personnes en situation irrégulière sur le territoire mahorais on attente de renouvellement de leur titre de séjour, on en arrive ainsi à des ruptures de couverture incompatible avec les objectifs poursuivis par le déploiement de la complémentaire santé solidaire à Mayotte, au-delà de cet article, Madame la Ministre, Monsieur le ministre, il y a donc nécessité d'augmenter les moyens financiers pour les soins à Mayotte et donner à nos concitoyennes et concitoyens la garantie pleine et entière de l'accès aux soins, je vous remet. Merci le mille. Trois du gouvernement, Madame la ministre. Monsieur le président, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, cet amendement vise à clarifier le régime applicable aux cotisations d'assurance-maladie due par les employeurs des fonctionnaires affectés à Mayotte. Merci, avis de la commission. Oui, monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, cet amendement, nous semble tout à fait cohérent et donc c'est un avis favorable, je vous remercie. C'est. Je mise aux voix, l'amendement mille trois avec du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour.

Qui est contre, il est adopté. à l'article 40 le sang trois Madame Gruny au nom de la commission. C'est un un amendement rédactionnel, monsieur le président. Oui du gouvernement favorable merci je mais on voit le centre de la commission avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Un nouvel amendement le CIV madame la rapporteure. C'est encore un amendement rédactionnel, monsieur le président. Merci avait du gouvernement favorable merci je mais on voit le CIV de la commission avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il est adopté, je mets aux voix, l'article 40 qui est pour, qui est contre, il est adopté. à l'article 40 bis Madame Jasmin. Merci monsieur le président, j'espère que ma voix, mieux que ce matin, la bonne santé financière de la branche accident de travail, maladies professionnelles après année ça augmente et permet un transfert de la branche de cette moi je vais la branche maladie, toutefois, il est important de mettre en oeuvre pour intensifier des actions de prévention tout mettre en oeuvre ont intensifié ses actions et améliorer les conditions de travail et particulièrement celle des femmes, des doté également les professionnels des équipements de sécurité et de protection et des potentiels Maurice des potentiels risques encourus j'attire, Madame la Ministre votre attention sur la situation des femmes dans tous les domaines et particulièrement dans la police nationale, l'association des femmes de la police dans la diversité, souhaite que des efforts soient faits en ce sens, c'est aussi le cas dans les différentes professions et particulièrement pour les professionnels de l'aide à la personne, je vous remercie et je vous remercie de votre attention à l'égard de ces personnes.

Merci je mais on voit le 106 de la commission avec accueil favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté, je mets aux voix le et l'article 40 quater est ainsi rédigé avant l'article 41 l'amendement de qui le défend. Alors Monsieur Hunault c'est un amendement de de Madame Goulet, monsieur le Président Madame Monsieur le ministre, il s'agit de lutter contre la fraude et notamment la fraude transfrontalière qui est connu et et massive et et de proposer que les organismes chargés d'optimiser la lutte contre les fraudes, notamment détachement dans le cadre contraignant fixé par laisser, j'ai eu soit mis en place ce jour merci. Merci, avis de la Commission, monsieur Savary. Oui, cet amendement vise à prévoir l'échange d'informations nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence auquel est est soumis le versement de certaines prestations entre la France et d'autres États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, c'est pas la fraude tanière doit effectivement être combattue avec détermination l'instauration d'un circuit d'échange d'informations entre États membres, devrait faire l'objet de travaux au niveau des institutions communautaires et découler d'un acte législatif européen et non pas national, donc c'est une demande de retrait ou d'avis défavorables. qui est éclairé continue à éclairer les décisions du gouvernement et les propositions que nous sommes amenés à reprendre, je pense qu'il s'agit avant tout ici d'un amendement d'appel pour appeler à ce que la coopération, la coordination entre les différents États s'agissant de la lutte contre la fraude, via la sécurité sociale ou les retraites se poursuivre en l'occurrence un système d'information, d'échanges d'informations mis en place le système d'échanges électroniques d'information sur la sécurité sociale, il continue à se mettre en place et son au Pérou rationalisation se renforce, mais donc en attendant c'est un une demande de retrait sinon défavorable. Merci retirer maintenu. Donc maintenu, allez je maintiens donc avec 2 avis défavorables de qui est pour.

Merci monsieur le président, madame le ministre, monsieur le ministre, il s'agit de donner des responsabilités aux présidents des tribunaux de commerce dans le domaine de la lutte contre la fraude, je vous remercie, commissions. écoutez à travers le texte d'amendement est satisfait, donc on peut le retirer. Gouvernement. Oui, ça faisait partie des propositions nombreuses du rapport et effectivement à l'article 41 de ce texte, nous donnons cette faculté de pour les organismes sociaux, d'obtenir des renseignements auprès des greffiers des tribunaux de commerce, donc : demande de retrait.

Commission. Oui, ça part d'une bonne intention pourrait effectivement penser que ces prestations doit va être mis sur un Livret A, mais comme après on peut faire des transferts d'un Livret A sur un autre compte, ça devient inopérant, c'est la raison pour laquelle j'ai donné un avis défavorable. Merci avait du ministre. Oui, d'abord, il n'est pas certain que ces dispositions et leur place dans une loi de financement de la Sécurité sociale sans lien Direct ensuite en termes opérationnels, je ne suis pas certain que ça changerait grand-chose on peut forcer à ce que les prestations soient versés sur un compte courant, rien, rien n'empêche ensuite de les verser sur un autre livret je pense que l'important et c'est une des avancées importantes c'est la disposition qui arrivent plus tard qui a été introduite à l'Assemblée par amendement du gouvernement qui est aussi une reprise d'une proposition de Madame Goulet, qui est de rendre obligatoire le versement des prestations sociales à l'avenir sur un compte, français ou européens, en excluant ainsi les comptes étrangers, ça me semble déjà être un un pas important.

nous demandons au niveau de la commission des affaires sociales, le retrait ou bien c'est un avis défavorable. Avis du Gouvernement Monsieur le Ministre. Oui, on m'a toujours appris qu'au Sénat, il fallait être très précoce ONU avec les demandes de rapport en l'occurrence il y a déjà beaucoup d'informations disponible sur ce sujet-là, notamment les travaux du le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, il a consolidé son rapport annuel relatif à la mobilité internationale, encore récemment, donc c'est une demande de retrait.

Oui, merci Monsieur le Président Madame Monsieur le Ministre, en fait Madame Goulet et m'a demandé de porter sa parole, vous l'avez dit, monsieur le Ministre, elle travaille depuis très longtemps sur les sujets de fraude et elle a une interrogation, moi la la question porte sur le lien entre les différents organismes sociaux et le fichier des étrangers en France, selon les dispositions de la loi, je cite, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité sociale du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionné au au présent code organise le contrôle du respect des conditions de résidence en France ce contrôle et chaque fois que possible, réalisée à partir des vérifications opérées par un autre organisme de Sécurité sociale, or elle constate que les contrôles en général ne sont pas faits, il n'y a pas de vérification systématique à l'entrée dans nos systèmes, ni en cours de route ni quand les gens perdent leur droit au maintien sur le territoire, elle donne l'exemple par exemple d'un étudiant Erasmus dont la carte n'est pas des désactivé en fin d'Erasmus c'est ainsi également que des personnes sans plus de droit au maintien sur le territoire conserve droit et carte vitale donc elle conseille elle recommande, ça fait partie des recommandations de faire une consultation systématique du Fichier âgé de rêve, elle a un amendement qui arrive un petit peu plus loin qui porte sur ce point aurait là une surprise très désagréable en consultant le budget asile immigration qui annonce, pour 28 millions à la création d'un nouveau dispositif qui remplacerait âgé de rêve dont la disparition est annoncée alors quelles sont les intentions du gouvernement est-ce que l'information est confirmée Si Madame Sollogoub l'amendement 1098 madame le héros. Merci monsieur le président, il s'agit de l'article 81 41 pardon qui renforce la lutte contre la fraude fiscale aux prestations sociales, notamment en rehaussant le plafond des pénalités financières qui peuvent être décidées par les fraudeurs qu'il s'agisse d'assurer de professionnels ou d'employeurs, si la fraude d'où qu'elle provienne doit évidemment être combattu il est dommage de concentrer les efforts sur l'une d'elles, uniquement quand les moyens mis dans la lutte contre l'évasion fiscale bien supérieur à la fraude sociale reste largement insuffisant pour rappel, cette dernière représente selon les suffrages entre Soissons des 100 milliards d'euros chaque année bien plus que les estimations, même les plus fortes de la fraude aux prestations sociales. écoutez cet article article 41 que l'amendement. Pose de supprimer prévoit des mesures importantes en matière de lutte contre les fraudes sociales et notamment l'attribution de pouvoirs de Cyber enquête sous pseudonyme aux agents de contrôle des organismes de protection sociale et aux organismes de l'inspection du travail, l'augmentation des plafonds de pénalités en cas de fraude à l'assurance maladie et encore la simplification de la procédure de mise en oeuvre d'une pénalité en cas de manquement ou de fraude dans les branches famille et vieillesse. D'après l'étude d'impact que ces dispositions permettrait de générer près de 50 millions d'euros de recettes supplémentaires chaque année et sur, au profit de la sécurité sociale, du reste, au delà de son coût, la fraude sociale mine le lien social et le consentement à la cotisation il importe donc de mobiliser tous les moyens ne disposition pour rechercher et sanctionner ces comportements inciviques, vous comprendrez bien que la commission a mis un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Oui, d'abord pour répondre à Madame Goulet via madame, le groupe qui s'est fait sa porte. Parole lui dire qu'on partage l'objectif de lutter contre ces fraudes que il y a des contrôles qui sont menées, s'agissant des personnes étrangères sur notre sol je, il peut y avoir des moments où il y a un petit délai ou un délai trop important, avant que les droits soient suspendus, vous avez donné un exemple sur un Erasmus, un exemple : pour une personne qui recevrait une se verraient délivrer une OQTF, il peut arriver qu'il y a un moment avant que les droits soient effectivement suspendu, or il faut rappeler le principe c'est quand vous êtes en situation irrégulière, vous n'avez pas de droits à prestations sociales sur notre sol et donc je pense que c'est effectivement dans les contrôles qui doivent se poursuivent et dans la célérité avec laquelle on est capable de de répondre qu'il faut avancer sur le remplacement âgé de rêve par année, oui, je vous le confirme l'objectif, c'est d'être plus efficace, c'est d'avoir un nouveau fichier élargie qui donne accès à des pièces nouvelles et qui donne accès aux documents eux- mêmes pour vérifier, par exemple, la validité des titres de séjour, donc l'objectif c'est d'être plus efficace, s'agissant des contrôles pour répondre à l'amendement porté par Madame Le Houerou évidemment avis défavorable puisqu'il viendrait supprimer cet article est un article très important s'agissant du renforcement de nos moyens de lutter contre la fraude sociale dans notre pays l'an dernier, c'est 1,5 milliards d'euros de fraude qui a été détecté, on souhaite aller plus loin, on parle en plus ici de fraude à réseau organisé et donc c'est extrêmement important qu'on dispose de moyens supplémentaires de levier supplémentaire, c'est ce que prévoit cet article notamment via ce dont on parlait tout à l'heure sur les échanges avec les tribunaux de commerce et les organismes de Sécurité sociale, mais aussi avec d'autres leviers, donc c'est important que cet article soit adoptée. Merci. Le mais où vois le 1098 avec 2 avis défavorable

alors cet amendement vise en fait à lutter contre les rendez-vous non honorés en dans la pratique de la médecine, ce sont des effectivement des des pratiques qui sont en en sans cesse augmentation alors à la fois le perturbe bon déroulement de du travail des médecins sur les territoires, quand même à la limite aussi le, la possibilité d'accéder à des patients à des rendez-vous puisque ils sont non honorées et du coup ça fait des plages vides et l'idée de pouvoir permettre de des pénalités dans des, dans des situations et des modalités fixées par décret, moi je pense qu'il faut avoir aucun tabou sur le sujet, ça c'est déjà la la première chose, l'enquête URPS en Île-de-France, médecin en Île-de-France a fait état en moyenne de 2 rendez-vous par jour non ses 28 millions de rendez-vous en France et parents qui ne sont pas honorés, actuellement, je pense que c'est pas acceptable d'autant quand on a des des difficultés d'accès aux soins pour chacun de nos concitoyens redire effectivement qu'un rendez-vous non honorés, c'est une consultation qui est perdu pour un autre patient, ça ne veut pas dire qu'il faut à pénaliser les patients qui sont empêchés, mais rien n'empêche un petit coup de fil pour effectivement expliquer expliquer qu'on ne peut pas aller le médecin peut se réorganiser et enfin il y a un vrai sujet sur les plateformes qui permettent des de des prises de deux 3 rendez-vous pour une même spécialité et je pense que là aussi il y a une vraie régulation à faire, alors je ne sais pas ce que va devenir cet amendement mais en tout cas je pense que c'est un un sujet pour lequel il faut vraiment Merci le. 156 n'est pas défendu, donc l'avis de la commission sur le 642 monsieur le rapporteur. Merci de de soulever un problème majeur quand même qui est ce ce nom rendez vous par contre, la solution préconisée me paraît pas la bonne hein, puisque c'est pas la la Caisse primaire d'assurance maladie ou les autres caisses qui ont un manque à gagner, hein, puisque le

Et ces personnes-là en conséquence. On ne peut pas infliger, demandez à la CPAM d'infliger une pénalité pour de l'argent qui ne doit pas toucher, c'est la raison pour laquelle l'avis est défavorable. C'est. Avis du gouvernement. le gouvernement partage le constat et le fait que c'est un vrai problème et ça remonte par ailleurs par les professionnels de santé eux-mêmes ces patients qui pose un lapin entre guillemets ou les no show comme on l'appelle parfois ce qui prend du temps médical, ce qui limite l'accès à l'offre de soins pour d'autres patients et et ce qui est véritablement insupportable pour des professionnels de santé qui le disent, ça peut arriver que sur une journée, il y ait un certain nombre de patients qui ne se présentent pas alors qu'ils ont pris rendez-vous donc on partage l'objectif qui est de lutter contre ce phénomène, la question c'est comment est-ce qu'on y arrive, la difficulté c'est que aujourd'hui, quand vous prenez rendez-vous, notamment via les plateformes vous ne communiquez pas votre numéro de Sécurité de sécurité sociale, donc c'est très difficile d'identifier la 2ème chose c'est qu'on travaille par ailleurs avec les plateformes pour répondre à ce que vous évoquiez sur la prise de plusieurs rendez-vous en simultané, il y a un gros travail qui est mené avec elles pour essayer de limiter ça mais donc il faut trouver un système qui permettrait effectivement de pénaliser ces comportements lorsqu'il se répète, on en parlait avec ma collègue Agnès Firmin Le Bodo, qui a des idées sur le sujet, donc moi ce que je peux vous proposer, c'est de retirer votre amendement qui a permis d'appeler l'attention sur ce sujet là, mais vous avez vu que notre attention est pleinement focalisés sur ce sujet et m'engager à ce qu'on poursuive les travaux peut être avec d'ailleurs vous pour trouver une solution dans les prochains textes. Merci. Je mais aux voix oui madame Guillotin. Je juste vous remercier pour la réponse, effectivement c'est un amendement d'appel, je vais le retirer mais pour autant je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille à des mesures qui soient efficaces sur un sujet qui est important.

mais vise à permettre aux directeurs de CPAM de prononcer un avertissement en cas d'inobservation des règles du code de la sécurité sociale et procède à divers ajustements. 2 rédactionnelle,

qui a eu un avis favorable et qu'on va vous proposer donc le gouvernement a un procédé aux modifications de forme demander. Et donc si mes collègues en sont d'accord, comme il n'avait pas été rectifié, nous avions émis un avis défavorable, mais compte tenu qu'il est maintenant rectifier nous émettons un avis favorable à cet amendement gouvernemental. Merci. Monsieur le rapporteur, le 987 donc du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est. Pour qui est contre, il est adopté. Ensuite, un amendement et un sous-amendement le 107 de la commission ben justement dont vous parliez à l'instant monsieur le rapporteur. Voilà voilà. Eh bien, comme on en a déjà parlé, on va dire que cet amendement est rédactionnel. Non, c'est pas le moment. Et le sous-amendement rédactionnel de. Oui c'est rédactionnelle pour coordonner avec le précédent, donc favorable à l'amendement de Monsieur Savary, sous réserve de l'adoption du sous-amendement. C'est, je commence par le sous-amendement

Alors l'article 41 renvoie à un article réglementaire du code général des impôts, qui n'a pas encore été créée donc cet amendement est rédactionnel infirmer ainsi d'éviter cette référence doublement problématique. Monsieur le Ministre favorable je mais on voit le 108 de la commission avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté, le 543 madame la présidente Gruny. Personne. monsieur le président, donc l'alinéa cinquante indique que les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis directement au procureur de la République, l'amendement ici vise à préciser que ces procès-verbaux sont également transmis, bien entendu, après accord du procureur à la personne concernée par la fraction dans un souci de respect de la procédure contradictoire mais aussi de transparence oh merci. Merci, Merci madame la présidente, cet amendement prévoit la transmission automatique à l'auteur d'une infraction des procès-verbaux établis en cas d'escroquerie et de faux et usage de faux, de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale dans la mesure où ils sont susceptibles de fonder des poursuites pénales engagées par le ministère public ces procès-verbaux présente un un caractère judiciaire aussi aux enfin de ne pas porter atteinte au déroulement de la procédure ou de ces opérations préliminaires sa transmission automatique sans autorisation préalable du parquet n'était pas envisageable, notre collègue Pascale Gruny ayant accepté de préciser qu'il ne pouvait être procédé à s'être cette transmission qu'avec l'accord du procureur, on peut émettre un avis favorable à cet amendement. Merci avait. Le gouvernement, Monsieur le Ministre. c'est ce sont des pièces qui sont des documents de nature judiciaire, une pièce de procédure pénale est couverte par le secret de de l'instruction, mais seul le procureur peut décider de sa transmission et donc pour ces raisons-là, on ne peut pas être favorable alors je je comprends que vous avez voulu préciser que c'est ce ce que le procureur peut décider de le faire, mais à ce moment-là, c'est déjà couvert par le droit actuel, donc je suis pas totalement convaincu par par l'amendement donc avis défavorable. Madame la présidente. la justice, elle ne donne pas les documents ou c'est très très compliqué, donc là il y a bien l'accord du procureur, sincèrement, parce qu'au moins on aura ça et le procureur peut peut dire non, donc ça, ça change pas à la fin pour lui mais en revanche, si c'est pas inscrit, ce sera un nom pour tous. Pas de changement, pas de changement, allez je mais on voit le 543 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Le 1099 madame le héros. Merci monsieur le Président, cet amendement est un amendement de repli qui tend à exclure du dispositif initialement prévu, les agents de l'inspection du travail, agences et les effectifs de la direction générale du travail sont en grande diminution depuis 2016 et 2018, ce sont 4 5 % de postes en moins d'agents de contrôle pourtant ces contrôles sont essentielles pour oeuvrer à la santé des travailleurs à l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise ou au respect du droit du travail, dans la mesure où il est urgent de donner davantage de moyens à l'inspection du travail pour qu'elle exerce des missions qui lui sont confiés, il ne semble pas opportun, ni nécessaire d'étendre la mission de contrôle en ligne des agents déjà en sous-effectif. Merci, Oui, alors effectivement, les moyens sont sont sûrement insuffisant donc vaut peut-être mieux modifier les pratiques. Je pense qu'à travers cet article, on arrive à modifier les pratiques en accordant des pouvoirs de Cyber enquête sous pseudonyme aux agents de compte. Trop de l'inspection du du du travail hein, c'est quand même une action de plus de lutte contre la fraude qui tient à coeur, Nathalie Goulet, mais la plupart des membres de cette commission, beaucoup plus largement, c'est une économie envisagée de 15 millions d'euros quand même sur le budget de la Sécurité Sociale donc je pense que il vaut mieux laisser cette, cette façon de de procéder au sein de ce Plfss donc avis défavorable de la commission. Avis du gouvernement. Oui, c'est très important de pouvoir doter ses ses agents de pouvoir de Cyber enquête effectivement pour être plus efficace dans la lutte contre la fraude, en l'occurrence les mécanismes de fraude qu'on vise ici, ce sont les usurpations d'identité de coordonnées bancaires, les activités fictives, les ressources non déclarés ou les réseaux transnationaux de recrutement, c'est important qu'il ait ces moyens supplémentaires et la caractérisation des infractions de travail illégal et plus complexe, je vois que vous votre sujet c'est de vérifier qu'on ne va pas déshabiller, entre guillemets, l'inspection du travail qui est chargé, évidemment, de missions de contrôle au profit de ces cyber enquêteurs, la réponse est évidemment non, d'abord, je veux dire que dans le PLF nous renforçons les Budgets de l'inspection du travail, avec 2 1000000 500000 euros supplémentaires pour des revalorisations indemnitaires des inspecteurs du travail pour renforcer l'attractivité de ce corps et la 2ème chose, c'est que nous visons une augmentation à 15 % des interventions des services de l'inspection du travail en matière de lutte contre le travail illégal et à 6 5 pour 100 en matière de fraude au détachement, vous voyez bien qu'on agit sur les 2 leviers ont d'autres, les agents de contrôle de pouvoir de Cyber enquête parce que c'est important pour démanteler ces nouvelles fraudes complexes mais on renforce aussi les moyens de l'inspection du travail pour ces missions : avis défavorable. Merci. Je mais voit le 1099 avec 2 avis défavorable qui est pour.

de suspendre les les droits sociaux des personnes visées par une OQTF, hein, une obligation de quitter le territoire français dont on parle beaucoup en ce moment, sauf évidemment en cas d'urgence je veux rappeler aussi que nous demandons depuis 3 ans une consultation obligatoire du fichier AG2R GDR bref avant l'ouverture des droits à prestation et que cette proposition, bien sûr, est en cohérence avec la condition de résidence régulière en France, je vous remercie. Merci avait là. Commission monsieur le rapporteur. Oui, cet amendement prévoit la suspension immédiate des droits à prestations sociales d'une personne faisant l'objet d'une OQTF. Il n'est en effet pas acceptable qu'un étranger séjourner en France de façon irrégulière et devant quitter le territoire, continuer à bénéficier de prestations, toutefois, le gouvernement a annoncé que c'est une mesure figurer au sein du projet de loi relatif à l'immigration, qui devrait être examiné depuis début 2023, il serait souhaitable que nous poursuivions nos réflexions dans cette attente de façon à perfectionner le dispositif. Et surtout à le sécuriser sur le plan juridique, ce que ne fait pas suffisamment cet amendement, c'est la raison pour laquelle la Commission demande hein. avis de de retrait, mais nous allons avoir la la position du gouvernement pour nous éclairer sur cette affaire-là. Merci monsieur le le le président : j'y vois là aussi un amendement d'appel puisque c'est d'ores et déjà le droit, le droit aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez bénéficier d'une prestation sociale que si vous résidez régulièrement en France c'est d'ailleurs l'exemple que je donnais tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit sur la question des contrôles et de l'application des règles, j'ai dit qu'il pouvait y avoir certains cas où les règles ne sont pas appliquées suffisamment fortement et suffisamment efficacement et j'ai donné l'exemple d'une personne qui se voit délivrer une obligation de quitter le territoire français et dont les droits ne sera pas suspendu immédiatement, ça fait partie des enjeux sur lesquels il faut qu'on progresse, ajouté cet amendement et cette obligation légale, alors que c'est déjà dans le droit n'est pas n'est pas nécessaire effectivement mon collègue Gérald Darmanin souhaite qu'on soit plus efficace en la matière, c'est-à-dire qu'on ait davantage de leviers de contrôle d'automatisation qui nous permettent vraiment de procéder à la levée de ces droits à prestations sociales, mais d'ores et déjà le droit prévoit que si on vous délivre une aucune obligation de quitter le territoire français, ça veut dire que vous ne résidait pas de manière régulière en France et donc vous n'avez plus le droit, vos prestations sociales donc demande de retrait sinon défavorable. Merci oui. Monsieur le président je maintiens l'amendement parce que je comprends l'argumentation m'être sincèrement, j'ai des doutes sur l'application réelle de ces dispositions et donc ça va encore mieux en le disant et en l'écrivant nettement lors de ce débat, je vous remercie. Merci monsieur non Monsieur mouillé. merci le président, nous allons bien entendu suivre notre rapporteur qui a des arguments clairs et qui explique que nous devons encore procéder à des travaux et que le la rédaction de cet amendement nécessite a en tout cas une sécurisation juridique, pardon monsieur le Ministre quand je vous entends, je pense qu'on ne vit pas sur la même planète parce que moi je suis dans mon département, l'ensemble des, des, des personnes qui reçoit cette obligation et aujourd'hui les droits continuent d'être versées, de la même façon, voire même les collectivités qui sont parfois qui accueille, là elle est on va continuent de percevoir pour outil de ces personnes, tous les droits possibles, alors je sais pas si c'est dans la loi mais concrètement dans l'application, ça n'existe pas, je nous avons des personnes qui sont dans des logements

Merci. Je vais donc mettre aux voix le 289 avec 2 avis négatifs qui est pour. Qui est contre Il n'est pas adopté alors après pour les votes suivant : si vous pouviez réellement levé la main, je comprends la gêne parfois de c'est d'être ni pour dit. Contres ni ailleurs, mais pour calculer de là-haut le le le côté je lève, je lève pas assez symbolique quand même hein, allez, il n'est pas adopté. 2 amendements identiques maintenant le 805 Madame Cohen. a été condamné le 15 septembre dernier pour traite d'être s'humains aggravée 26 femmes de ménage ukrainienne sans-papiers ont été reconnus victimes de leur ex-employeur de les avoir surexploité dans les conditions indignes de travail dissimulé constitue une double honte honte sociale et humaine en ce qui l'entraîne des conditions de vie indignes honte fiscale en ce qu'ils vole la collectivité nationale, qui a fait le choix politique d'une mutualisation, son système de protection sociale, le contrat de travail consacrent la relation asymétrique de pouvoir entre l'employeur et l'employé son respect la protection minimale du à chaque travailleur son absence, son illégalité ou le manque de toutes obligations afférentes, tels que le versement des cotisations patronales entraîne donc une sanction bien légitime, le Conseil constitutionnel a même reconnu que la lutte contre la fraude revêtaient le caractère d'une exigence constitutionnelle en 2019, une note confidentielle de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale à cause que le journal Les Échos avaient pu consulter soulignait que le travail dissimulé, était responsable d'un manque à gagner, compris entre 5 2 et 6 5 milliards, soit entre 1 7 et de un pour 100 des cotisations, c'est que ces conclusions appellent un volontarisme accru pour une pratique utilisée autant de la part de grandes aux entreprises comme Ryanair année cette année à payer près de 4 à 5 milliards à l'Urssaf ou c'est 65 entreprises du Lot, qui ont dû s'acquitter de 250232 euros au même organisme la probité ne s'achète pas, mais les dettes que l'on a auprès de la collectivité si nous proposons donc d'augmenter les sanctions à l'égard de ces délinquants récidivistes qui attendent, moralement, humainement et financièrement qui a atteinte qui ont une atteinte à nos systèmes, je vais y arriver social en voulant aller vite, on s'embrouille. Merci. Madame Cohen, mais on avait tous compris l'amendement cent identiques, madame le héros. Oui merci, donc cet amendement répond en évidemment à une grande préoccupation de notre part, mais également à une préoccupation de la Cour des comptes qui pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales, nous estimons que ce que le volontarisme affiché du gouvernement devrait se concentrer sur la fraude aux cotisations sociales patronales telles qu'elles ont été des décrite par ma collègue la fraude patronale aux cotisations sociales coûtent chaque année près de 8 milliards d'euros aux caisses de Sécurité sociale, soit autant que les économies attendues par Monsieur Macron pour sa réforme des retraites, sur ce montant, à peine plus de 700 millions d'euros sont merci. Merci avec. Oui, monsieur le président, cet amendement donc à bord le le le les récidives de travail dissimulé. En majorant les, les, les sommes à redresser en les doublant selon la constatation des infractions mais l'arsenal de sanctions actuellement implique applicable nous paraît suffisamment dissuasif, d'autant que s'y ajoutent des mesures d'annulation des exonérations ou réductions de cotisations sociales dont bénéficient l'auteur de l'infraction que l'article 6, tend à renforcer pour les donneurs d'ordre récidiviste et qu'il y a également des sanctions pénales et des sanctions administratif, donc l'arsenal étant là. Nous avons donné un avis défavorable à la proposition faite par nos. Collègues avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, vous voulez lutter davantage contre le travail dissimulé et on partage évidemment cet objectif quand on parle de lutter contre la fraude sociale, on parle pas uniquement de lutter contre la fraude de celui qui touche du Mans, une prestation, on parle aussi de lutter contre le travail informel le travail 18 dissimulé des réseaux qui sont en débat organisé de la fraude aux cotisations sociales par les entreprises, vous avez raison, c'est important de le rappeler, c'est d'ailleurs l'an dernier 800 millions d'euros qui ont été recouvrés au titre du travail informel en forte augmentation, moi j'ai vraiment salué le travail de nos services pour augmenter les contrôles, être plus efficace dans les contrôles et pouvoir recouvrer effectivement en cas de de de fraude manifeste le problème qui a, avec votre amendement c'est que proposait de majorer les sanctions existantes mais en le faisant et je pense que ça n'est pas votre objectif vous écraser en tout cas vous supprimez un autre dispositif de sanctions qui est la suppression des exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises lorsqu'elles fraude quand une entreprise on détecte une fraude manifeste est majeur, on lui supprime le droit aux exonérations de cotisations sociales et je sais en plus que sur vos bancs, vous êtes assez opposées d'une manière générale à ces exonérations de cotisations sociales, donc j'imagine que ça n'est pas votre intention que de leur permettent de continuer à en bénéficier, d'autant plus quand elle fraude en l'occurrence, en 2021 c'est 21 millions d'euros qui ont été. Récupéré par les Urssaf à ce titre-là, et donc votre amendement supprimerait cette possibilité je rappelle, par ailleurs, et le rapporteur le rapporteur la fait que nous avons déjà un dispositif de redressement avec des majorations complémentaires qui existe et donc in fine et votre amendement reviendrait à restreindre les possibilités de redressement dont nous disposons, je ne pense pas que c'est l'objectif donc : demande de retrait sinon défavorable. Très bien. Je mais on voit le 805 et le 1100 identique avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre, ils sont rejetés. Monsieur nos j'imagine pour le sept oui, vous imaginez bien, monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, différents rapports, notamment celui de la Cour des comptes ou encore les rapports de mesdames Granjean écoulé, ont souligné les fraudes en en matière de retraites versées à l'étranger, et donc il s'agit de contrôler l'existence des bénéficiaires, il y a pas qu'en matière de vote hein, qu'il faut contrôler l'existence des bénéficiaires pour ce qui concerne aussi le versement des retraites à l'étranger, je vous remercie. S'il avait. La commission, monsieur le rapporteur. Madame Goulet va être. Puisque cet amendement vise à rétablir les dispositions de l'article 83 de la loi de finances pour 2013 qui prévoit le contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite servies par un régime Français établis à l'étranger en fait l'article 104 104 pardon. De cette loi de financement pour 2021 à actualiser les dispositions qui figurent désormais aux articles sortait un 24 3 du code de la sécurité sociale, tout en permettant aux retraités d'apporter la preuve de leur existence, par le biais de données biométriques en conséquence, l'amendement est satisfait c'est la raison pour laquelle je pense que vous pouvez le retirer. Avait du gouvernement. André la de feuilles. Oui effectivement en droit, s'est satisfait, mais je pense que ça vise à attirer notre attention sur les phénomènes de fraude aux prestations sociales, en l'occurrence ici aux retraites pour des personnes qui seraient décédés qui n'existerait plus, entre guillemets, et dont la retraite continuera à être perçu par des personnes de l'entourage, évidemment que c'est une préoccupation qu'on a, s'agissant de l'ensemble des allocations et prestations sociales que de limiter au maximum ce type de fraude, c'est la raison pour laquelle un des articles qui arrive après est issu d'un amendement que j'ai porté à l'Assemblée nationale et il vise maintenant à conditionner le versement d'allocations sociales à un compte bancaire français ou européen, parce que le fait de passer par un compte français ou européen et quand même une très un très bon moyen de vérifier l'existence de la personne, les banques le font, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sur les retraites, parce que la retraite n'est pas une prestation soumise à condition de résidence pouvait avoir travaillé toute votre vie en France bénéficie à ce titre d'une retraite, mais décidé prendre votre retraite ailleurs dans un autre pays et vous l'avoir versé sur un compte étranger, donc il faut une politique plus ciblée pour contrôler effectivement l'existence des bénéficiaires de d'allocation retraite à l'étranger, on sait qu'il y a certains pays avec lesquels il y a, voilà plus d'enjeu, hein, je vais je je je n'apprends rien ici, c'était dans les rapports que vous avez évoquées notamment certains pays du Maghreb, donc je pense que, indépendamment du droit qui est déjà satisfait, en l'occurrence l'enjeu, c'est la question du contrôle, je viens de détacher il y a quelques mois, des agents dans nos consulats dans les pays concernés pour qu'ils puissent procéder à des contrôles en convoquant des personnes pour lesquelles nous avons des doutes voilà et je pense que ça fait partie des leviers qui nous permettent d'être plus efficace dans nos contrôles, nous demande de retrait sinon défavorable. Merci Monsieur Viénot,

merci avec de la commission. ou dans la zone européenne élargie, les prestations sociales soumise à condition de résidence en France il serait évidemment préférable d'appliquer cette mesure, le plus rapidement possible, c'est la raison pour laquelle Nathalie Goulet propose de l'appliquer dès le 1er juillet 2023 et non pas attendre 2024 donc nous sollicitons l'avis du gouvernement sur cette proposition C'est une disposition qui a beaucoup fait parler, effectivement, c'était une mesure qui était proposée par Madame Goulet dans sa proposition de loi, je crois que c'était l'article 14 que j'ai reprise dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, en première lecture à l'Assemblée nationale et j'ai porté un amendement du gouvernement pour conditionner le versement des prestations sociales soumise à condition de résidence à un compte bancaire français ou européen et ça a été très commentés puisqu'ensuite, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de commentaires sur Internet, les réseaux sociaux que j'ai regardé l'écrasante majorité évidemment des personnes a été favorable à cette mesure et la soutenait, mais un commentaire qui revenait le plus, c'est pourquoi attendre un an puisque on a prévu dans le texte, effectivement, que ça soit au 1er janvier 2024 on avait effectivement prévu ce délai d'un an, d'abord pour être sûr que les caisses de Sécurité sociale soit prête pour mettre en place cette obligation, ça c'est la première chose et ensuite pour qu'il y a un délai de prévenance pour des personnes qui bénéficierait effectivement de ses prestations sociales sur un compte étranger qu'elles aient le temps de s'ouvrir un compte, français ou européen, depuis l'adoption du Plfss en première lecture à l'Assemblée, nous avons échangé avec les caisses de Sécurité sociale qui nous ont dit qu'elle pourrait être prête plus tôt, je pense par ailleurs que nos concitoyens ou les personnes concernées ont eu vent de cette mesure et l'ont entendu donc je donne un avis de sagesse à cet amendement qui prévoit d'avancer de 6 mois et ça veut dire mettre en oeuvre cette obligation 1er juillet 2023 en lieu et place du 1er janvier 2024. Avis de la commission sur le coup. Alors. C'est le ministre compte tenu de ces éléments, je pense qu'il est intéressant de voter cet amendement pour fixer la date le plus tôt possible. Donc, avis favorable Monsieur valant. Et comme j'avais effectivement rapporté sur la PPL de madame Boulay je me réjouis, monsieur le Ministre, que vous ayez effectivement repris et que vous repreniez aussi cet amendement parce que ça c'est vrai que plus tôt sera le mieux pour éviter effectivement les fraudes, donc je me réjouis, mais je j'en profite pour vous poser une question : puisque vous n'étiez pas là lors de la discussion générale, c'est sûr, les estimations que nous avons sollicité, notamment auprès des caisses, et en particulier auprès de la caisse d'assurance maladie et que nous attends, nous attendons, et j'espère que vous pourrez accélérer le procès la procédure pour que nous puissions avoir on l'espérait pour ce PLFSS nous puissions avoir des estimations.

Ce que je remarque quand même c'est que vous avez, vous mettez beaucoup de moyens pour vous diligentée beaucoup de moyens quoi il s'agit effectivement de ce qu'on appelle la fraude sociale aux prestations et c'est très bien, mais je vous rappelle quand même d'ailleurs on devrait toujours préciser de quelles fraudes sociales on parle la fraude sociale aux cotisations et 9 fois plus importante ma collègue, il a dit son rendement est est plus que ridicule, donc Monsieur le Ministre quand est-ce que vous allez diligentée les moyens à la hauteur de la fraude sociale aux cotisations. Merci, attendez, attendez, vous avez d'abord Monsieur lévriers vous allez pas vouloir répondre avant. Merci monsieur le président, juste une toute petite remarque on, on peut imaginer que nombre de ces retraites sont des petites retraites et que donc, nombre des les personnes qui les seront peut-être des difficultés sur tout ce qui est documents administratifs, donc je trouve que le délai de 6 mois et très bien excellent, à une condition, c'est que la communication autour, se passe très bien aussi pour ne pas pénaliser des gens de bonne foi qui n'arrivera pas à s'informer sur ce sujet, merci. merci Monsieur le Président, mais pour vous répondre : oui on a besoin de pouvoir davantage documenté, ce dont on parle, il y a aujourd'hui multitude de rapports et d'études qui ont été réalisées, vous avez des études qui ont été réalisées par l'assurance maladie s'agissant des professionnels de santé, vous en avez qui ont été réalisées par la CNAV, s'agissant de à l'ASPA ou du minimum vieillesse, vous avez des rapports de la Cour des comptes, vous avez des rapports sénatoriaux, moi ce que je souhaite, c'est mettre en place un un comité indépendant d'évaluation de la fraude aux prestations sociales, je précise, hein, ça, ce sera pas une nouvelle, un nouveau comité avec des moyens entre guillemets une main, et cetera, on va, on mettra à disposition les moyens des administrations de Bercy et de la sécurité sociale auquel on veut associer des parlementaires, des personnalités qualifiées pour être capable d'être plus efficace et exhaustif sur ce qu'on est capable de de mesurer de cette fraude aux prestations sociales, donc ça c'est un un chantier qu'on va lancer dans les prochaines semaines, les prochains mois pour vous répondre madame la sénatrice. évidemment, moi je ne fais pas de concurrence ou je je je je ne je n'oppose pas les fraudes, enfin je je ne considère pas qu'il y a un type de fraude qu'il faut davantage poursuivent que les autres toute fraude est inacceptable frauder c'est voler c'est miné le pacte républicain et le pacte social, donc toutes les fraudes, doivent faire l'objet de la même intensité dans la lutte qui est menée par les pouvoirs publics et je peux vous dire que mes services à Bercy, s'agissant de la fraude fiscale sont particulièrement mobilisés l'an dernier, montant record de droits notifiés en matière de fraude fiscale, plus de 13 milliards d'euros 11 milliards d'euros recouvrer on va de record en record, on renforce nos moyens notamment aussi avec l'apport du numérique aujourd'hui vous avez plus de 50 % des contrôles fiscaux qui sont guidées orientées par l'Intelligence artificielle grâce à des algorithmes qui nous permettre de détecter des indices et qui permettent ensuite de guider les agents vers le contrôle des personnes ou des estime qu'elles sont, qu'il est plus probable qu'elle réalise des fraudes et sur la fraude aux cotisations sociales au travail dissimulé, on a vu tout à l'heure j'ai rappelé l'ambition qui est la nôtre, les moyens dont on dispose donc, vraiment, de ce point de vue là toutes les fraudes doivent être convaincus combattu avec vigueur.

il me paraît indispensable parce que moi je n'ai pas compris comment une application au 1er janvier 2024 avait un impact sur la LFSS 2023 donc, enfin, je ne vais jamais vu ça, donc voilà donc évidemment qu'il vaut mieux mettre la date en 2023 pour éviter une éventuelle censure bon et puis, pardon monsieur le président, mais je je réagis quand même au promet aux propos du du du ministre parce que oui on et frauder c'est voler, bon, d'accord oui sauter la barrière du métro c'est frauder c'est voler tout n'entraîne pas la même mobilisation et ne doit pas entraîner la même mobilisation la fraude des employeurs, la fraude patronale. C'est comme l'évasion fiscale, ce sont des fraudes qui sont massives et qui déstructure profondément une société la fraude d'un individu au prestation, ça doit être sanctionné, bien sûr, mais la fraude d'un individu aux prestations, c'est un individu point la fraude d'organisation l'évasion fiscale des multinationales qui ne payent pas l'impôt en France des dizaines, des centaines de milliards qui échappent aux sociétés à nos sociétés, ce sont des puissants Fasseur de facteur de déstructuration de la société et pardon mais dans vos engagements, on vous entend beaucoup plus sur la fraude aux cotisent aux prestations que sur cette fraude-là, bon, on note que vous êtes venus pour ce PLFSS en séance avec nous pour parler de la fraude malheureusement vous a pas vu au moment des recettes de cette discussion de comment on crée des recettes pour notre sécurité sociale, pour les prix pour les prestations qui sont versées dans notre pays pour la santé, pour la vieille bon vous êtes venus pour parler de la fraude et à 80 % de la fraude aux prestations, voilà c'est tout. Je je vais redonner la par le ministre des je, je voudrais qu'on en reste à l'article

c'est pas l'article 41 bis, mais Monsieur le Ministre, allez-y. pour le projet de loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale, je n'ai pas encore le don d'ubiquité, ni d'hologrammes qui me permettrait d'être présent dans les 2 chambres en même temps, mais je crois être 13 à disposition du Sénat régulièrement, j'étais aussi auditionné par la commission des affaires sociales récemment. Sur ces sujets, la 2ème, chose que je veux dire, c'est que si je vous écoute, vous devriez vous réjouir et félicité ce gouvernement, ce président de la République, qui ont fait sauter le verrou de Bercy en 2018 félicité ce gouvernement, ce président de la République qui aligne les grandes entreprises les unes après les autres pour des mécanismes d'optimisation fiscale, cet été, mes services ont mis une amende record à Mac Donald, 1 milliard 200 millions d'euros, 200 millions d'euros pour Mac Donald pour des mécanismes d'optimisation fiscale encore récemment pour de l'accompagnement qui était réalisée par le Crédit Suisse sur l'optimisation fiscale aussi 300 millions d'euros d'amende qui ont été notifiés, des, des amendes qui sont prononcées et notamment parce qu'on a des nouveaux leviers via la loi de lutte contre la fraude en 2018 qui sont record et je trouve que vous devriez plutôt salué reconnaître cette action que de considérer que rien n'est fait, puisque c'est absolument pas vrai. Merci. Alors est-ce que cet amendement est maintenu ou pas. Monsieur et nous, il est maintenu, alors je le mets aux voix je ah au bout du bout, on ne sait plus avec la vie quoi, d'ailleurs, monsieur le rapporteur, appelez-nous, après tout ça à l'avis de la commission est favorable, l'avis du gouvernement est favorable sagesse sagesse allez le 152 donc, avec un avis favorable de la commission sagesse du gouvernement qui est pour. Toc qui est contre, ben voilà, il est adopté l'article 41 bis nouveau je le mets aux voix qui est pour. Qui est contre. Il est adopté à l'article 42 Madame Sollogoub. Oui, merci Monsieur le Président Madame Monsieur le Ministre, je propose de supprimer cet article parce que il ajoute des pénalités financières allant compte des professionnels de santé, en cas de fraude ainsi que des possibilités de mise hors convention alors qu'il existe déjà une procédure de pénalité financière et une procédure de déconventionnement qu'il suffit en fait d'utiliser,

que cet amendement tend à supprimer l'article 42 cet article permet notamment d'de la procédure de déconventionnement d'urgence applicables aux professionnels de santé, de l'étendre aux pharmaciens d'officine distribuait auteur de produits et prestations de santé et aux entreprises de transport sanitaire et de taxis conventionnés, ces dispositions permettent pourtant de faire cesser les comportements fautifs d'endetter les raccourcis, tout en étant très encadré, ces nouvelles dispositions, les directeurs de CPAM ne peuvent ainsi prononcé le déconventionnement d'urgence que lorsqu'un professionnel de santé, viole de manière particulièrement grave, les engagements prévus par la convention ou qu'ils résultent d'une telle violation un préjudice financier pour la CPAM et après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations, la durée du déconventionnement ne peut alors excéder 6 mois pendant lesquels le directeur de la CPAM doit engager la procédure normale de déconventionnement le professionnel pantoute demander à être entendu et présenter des observations écrites, alors maintenant, compte tenu de la persistance d'un pertinence de ce dispositif au regard de l'objectif de lutte contre la fraude sociale nous émettons un avis défavorable pour supprimer cette. Merci madame la ministre. Monsieur le président, dans la masse, sénatrice, je vais pas redire ce que vient d'expliquer à monsieur le rapporteur, mais vous proposez de supprimer cet article supprimé cet article-là, ça veut dire se supprimer une opportunité parce que je le dit cet article élargit le nombre de professionnels qui seraient soumis à des sanctions en cas de fraude, nous partageons le même motif de la lutte contre la fraude supprimer cet article c'est se passer d'une liste de professionnels élargie, pour lequel nous pourrions lutter contre la fraude, donc nous émettons un avis défavorable. Retirez retirez je mais on voit l'article 42 qui est pour. Qui est contre, il est adopté. à l'article 43 2 amendements identiques d'abord le 800

de mettre un coup de frein aux plateformes commerciales de téléconsultation tout en envoyant un message de fermeté face aux abus assimiler les salariés en arrêt de travail à des fraudeurs est inacceptable alors que, d'une part, les arrêts maladie sont accordés par les médecins eux-mêmes et non par les salariés, d'autre part, les salariés qui ont recours à la télé téléconsultation font partie, faut-il le rappeler des 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant et puis parfois il y a ceux et celles qui ont un médecin traitant, mais qui ne peut pas les recevoir appeler après plus plusieurs jours parce que je vous rappelle quand même que nous sommes dans des déserts médicaux donc dérembourser les, les arrêts de travail, comme le propose le gouvernement ou limiter la durée des tas, des arrêts de travail, comme le propose la majorité sénatoriale, remet en cause le droit à l'accès aux soins au médecin généraliste et remet en cause l'indemnisation maladie pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article, merci.

le médecin non, on ne le sous. Nous sommes de rien mais par contre, quand même, on perpétue la politique du soupçon, parce que ces dispositions se fonde un peu sur le fantasme d'un travailleur cherchant à multiplier les arrêts maladie de façon frauduleuse quand même via la télé consultation rappelons-le quand même, il y a 13 millions 13 millions d'arrêts maladie prescrits chaque année 600000 leçon en consultations et seulement 100000 sont, je le répète, 13 millions ne l'ne l'ont pas été par le médecin traitant, donc nous allons passer dix minutes sur ce petit nombre cette disposition s'attaque donc à une extrême minorité sont jamais les raisons pour lesquelles certaines personnes passent par la télé consultation pour les arrêts maladie, j'en reviens pas sur le fait, c'est tout en y revenant que 6 millions de personnes n'ont pas de médecin traitant que 3 millions d'entre elles n'en ont jamais eu et qu'on compte en moyenne 10 jours d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un médecin, alors que le délai pour envoyer son attestation attestation à la sécurité sociale et de 48 heures les populations en grande précarité ou vivant dans une zone sous-dense, bien qu'on me dit que c'est pas peu plus vont de nouveau souffrir de cet effet de loupe, hein, c'est un effet de loupe donc après avoir encouragé le recours à la télé, consultation ce recul sur les arrêts maladie par le gouvernement porte atteinte à fortiori dans certains territoires ou pour une certaine population à la capacité des travailleurs à préserver leur santé pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de l'article 43 43 effectivement quelque part. C'est l'arrêt de travail qui est un peu dans le quand même fragilisé par cet article. Merci. Madame la rapporteure. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement et est contraire à la position de la commission, il est important de veiller à limiter les abus en matière de téléconsultation et de prescriptions d'arrêts de travail ainsi veiller au bon usage des dépenses d'assurance-maladie, j'assiste, comme je l'ai fait en en commission sur le fait que la prise en charge d'arrêt de travail en consultation physique bien sûr n'est nullement remis en cause par cet article dans cet un avis défavorable à ces amendements de suppression.

un médecin traitant, et que 75 % de ces arrêts de travail non non été accompagnés d'aucune ordonnance que ce soit de médicaments ou que ce soit d'un acte de kiné, par exemple, donc il nous paraît important de redire à quel point la téléconsultation et le développement de la téléconsultation et majeur pour répondre aux besoins de santé mais que lutter contre la fraude est aussi est aussi un acte important, comme l'a dit à Madame, la rapporteure, donc, c'est pourquoi nous mettant un avis défavorable à sa maman. Merci de ne pas vous interpeller en séance je mais on voit ces deux amendements identiques avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Ils sont rejetés. Allez, allez, le 207 Madame Sollogoub. merci Monsieur le Président Madame Monsieur le Ministre, je reviens sur ce sujet qui est réellement essentiel sur nos territoires, enfin je je rejoins mes collègues, on rencontre tous les jours maintenant des gens qui sont absolument désespéré parce que c'est pas qu'ils choisissent pas leur médecin, c'est qu'ils ne trouvent pas de médecin traitant et quand éventuellement en désespoir de cause, soit ils renoncent aux soins, soit ils ont vraiment besoin de s'arrêter pour quelques jours, ils font quand même appel à une téléconsultation alors on en a échangé, monsieur le ministre, en commission, vous avez eu la la gentillesse de me répondre, vous avez dit on, on voit une espèce de dérive qui est en train de, pour l'instant, qui ne représente pas des sommes colossales, mais on voudrait stopper le phénomène avant que ça monte en puissance, malgré tout, c'est vrai que, plutôt que de pénaliser qu'y ait des gens qui sont déjà à la peine est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution intermédiaire, par exemple, imaginer un dispositif d'agrément pour le médecin qui pourrait pour voilà qui fasse preuve de manière à ce que lui aussi porte une responsabilité parce que c'est vrai qu'on a vu ça été médiatisé, les arrêts maladie en 3 minutes, de gens qui ne sont jamais vu c'est : c'est trop facile, mais est-ce qu'on peut pas plutôt que de pénaliser le patient, trouver un dispositif intermédiaire qui met aussi en jeu la responsabilité du médecin et puis qui évite de de d'un d'infliger la double peine aux patients qui n'ont pas médecin traitant. monsieur le président, ben c'est un amendement de repli qui propose que la suppression de l'indemnisation des arrêts de travail prescrits dans le cadre d'une téléconsultation ne vise pas les consultations effectuées dans le cas où le médecin traitant est absent ou et où ces consultations sont assurées alors par un médecin remplaçant il n'y a pas de problème, mais un médecin collaborateurs pour le serait visé par cet article si c'est ici c'est pas exclu, il est en effet absurde de pénaliser les patients dont le médecin traitant est absent ou indice ou indisponibles et serait abusif d'en conclure à une quelconque volonté de fraude de la part de l'assurer cette disposition est par ailleurs potentiellement compatible avec les diverses stratégies permettant de libérer du temps médical en zones sous-denses, en permettant aux médecins de transmettre la consultation à son collaborateur, le cas échéant, de plus, il appartient au médecin traitant, absent de veiller à ce que son remplaçant et bien d'accès à l'historique des consultations réalisées par le médecin traitant et soit en mesure d'apprécier la nécessité délivrer un arrêt de travail, ainsi il n'existe a priori aucune raison qui viserait à empêcher que les dispositions de l'article 43 soit complété en permettant aux remplaçants, et j'insiste, aux collaborateurs de médecin traitant de constater l'incapacité physique maintenant un arrêt de travail en télé consultation. Avis de la commission, alors rapporteur. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, alors sur, sur l'amendement 207 j'entends bien les préoccupations de de nos collègues concernant les possibilités d'accès à un médecin rapidement je vois malheureusement dans ces amendements, une sorte de de renoncement, comme si la consultation devenait l'offre de soins par défaut dans les zones sous-denses, ce qui me ce qui me semble aussi préoccupant sur le fond, je l'ai dit en commission, le dispositif ne sont pas opérationnels, comment prévoir qu'il y aura des médecins agréés en nombre suffisant, et ce tous les jours pour assurer les téléconsultations pouvant donner le droit à un arrêt de travail surtout l'amendement laisse ça à penser qu'il faudrait agréé des médecins pour s'assurer de leur éthique et de la justification de leur prescription, ce qui est un petit peu embêtant quand même, enfin, je leur dis à nouveau pour rappel Arctique maintient la prise en charge, or, médecin traitant à tout médecin vu récemment ou à toute consultation présidentielle, donc on est bien là sur un article qui souhaitent à à éviter les dérives, hein, d'arrêt de travail un peu trop complaisantes et les consultations, donc l'avis de la commission est défavorable sur l'amendement 945 donc, là aussi, je l'avais dit en commission cet amendement semble peu opérationnel et sans doute pour partie satisfaits en effet leur en téléconsultation le médecin titulaire sont bien inscrit sur l'acte même lorsqu'il est remplacé, donc ça fonctionne pour le médecin remplaçant la ministre pourra certainement confirmé ce point et concernant le médecin collaborateur, cela me semble peut-être plus difficile à à mettre en oeuvre, là encore, la consultation physique rend la prise en charge possible or médecin traitant et hors médecin vu récemment, donc ça l'avis défavorable de la commission. Merci à vide, la Ministre sur les deux amendements.

garantit en rien la possibilité d'avoir accès aux médecins, en plus, il crée sans doute une rupture d'égalité, donc là c'est encore sans doute en effet que vous ne souhaitiez pas atteindre, je le redis, il ne s'agit pas d'interdire les arrêts de travail, mais bien de lutter contre les abus, c'est bien la volonté que nous partageons tous, donc un avis défavorable, notamment pour la rupture d'égalité qu'il créerait entre nos concitoyens sur l'amendement 945 de Madame Poncet Monge, l'amendement est déjà satisfait parce que la possibilité pour un médecin remplaçant de pouvoir prescrire existe déjà, donc un retrait sinon avis défavorable et puis vous dire que, bien sûr, nous avons aussi ouvert la possibilité si le médecin traitant n'est pas disponible que le mais ce que le patient qui a vu un médecin de moins d'un an, puisse faire la télé consultation et donc nous avons élargi à ce dispositif pour pouvoir faire rembourser sa télé consultation.

les arrêts de travail prescrits par les spécialistes qui soit chirurgien ou parfois dans d'autres spécialités qui voit les patients et qui donne des arrêts de travail très court, en souhaitant que le le patient faire prolonger son arrêt de travail qui est tout à fait justifiée par le médecin traitant, or actuellement avec le problème d'encombrement des consultations chez chez les médecins, il y a des problèmes de de prise de rendez-vous et on voit des patients qui sont en bout d'arrêt de travail pour quelque chose qui justifie pleinement une prolongation

pouvoir non pas voir en rapport, puisque c'est pour ça, mais vraiment alerter ou que chacun prenne ses responsabilités et ne provoque pas des consultations inutiles simplement pour des démarches administratives. Merci. Je mets donc aux voix le 207 avec deux.

complaisance mais qu'est-ce que ça veut dire mais mais mais c'est grave de dire ça, même en téléconsultation, c'est un médecin qui est derrière l'écran

bon je suis malade, quelques fois le lundi, j'ai un rendez vous le jeudi ou le vendredi ou, au mieux, le mercredi soir, non mais je suis bien obligé de faire une téléconsultation je prends mon cas, mais c'est le cas de, de, de, de centaines de personnes dans mon département et donc moi je connais des gens qui passent par une téléconsultation parce qu'ils sont malades, on leur donne un arrêt de maladie, et je n'ai pas l'impression que c'est de la complaisance, mais j'ai quand même l'impression que, voilà, il faut réagir et et quand on a un patron, on est bien obligé de lui donner un arrêt de maladie, quand on est malade ou alors on fait comment va malade au boulot, enfin moi je suis je trouve vos propos scandaleux. Bien. Enfin pas bien sûr ce que vous trouvez scandaleux mais bien. Et vous avez largement dépassé la minute mais bon, vous aviez droit de vous aviez droit de Madame Cohen, ne vous inquiétez de rien, allez,

allons-y Monsieur. Mais pour pour une fois, monsieur le président, je ne vais pas faire de corporatisme, on me le reproche suffisamment pour ne pas en faire cette fois-ci, vous avez juste aller dans le sens qui a été dit par Madame pour ce polie pour signaler par exemple que dans ma région, la Provence-Alpes-Côte d'Azur dans un grand hôpital que je ne nommerai pas entre le mois de mai, au mois de septembre, le vendredi Monsieur le Ministre arrive entre 1000 et 1200 arrêt de travail pour trois jours. Bien voilà chacun en fera son miel mais je n'irai pas plus loin, je mais aux voix Pep et merci tu le vote je mais on voit donc le 207 avec 2 avis négatifs qui est pour. Oui, Madame Sollogoub, c'est le vôtre alors voter le oui qui est contre, voilà il est rejeté le 945 2 avis négatifs. Oui, qui est contre, il est également rejeté le 222 Monsieur De Gaulle. Alors, c'est le seul président, cet amendement vise à engager les médecins à orienter systématiquement des patients qui été les consulte vers une solution pour pouvoir bénéficier d'une consultation rapide lorsque l'état de santé, nécessite, afin de ne pas être pénalisés par la suppression des indemnités journalières, lorsqu'un arrêt de travail est justifiée. Merci. Ah oui, la rapporteure. Alors cet amendement décrit de manière détaillée ce que peut faire un médecin qui reçoit un patient téléconsultation la loi n'a pas à écrire les protocoles de soins ni à dire aux médecins qu'ils peuvent orienter leurs patients vers des soins ou examens complémentaires, donc c'est un avis défavorable de la commission. Ah oui du gouvernement. Un avis défavorable, parce que vous vous souhaitez engager les médecins télé consulter à orienter systématiquement les personnes vers une solution pour pouvoir bénéficier d'une consultation en physique aux arguments sont paradoxaux parce qu'il suppose que le délai d'obtention d'un rendez-vous médical physique serait plus rapide après une téléconsultation rien ne le garantit, et en plus la consultation physique doublera avec une téléconsultation, donc la sécurité sociale prendrait en charge de consultation pour le même objet, donc nous mettons un avis défavorable. Merci monsieur de colle. J'ai pour habitude de graver dans le marbre pour que ce soit plus simple, mais dans cette situation, je vais le retirer. Merci. 3 amendements en discussion commune le 946 madame pour Oui merci monsieur le président, alors il s'agit quand même de diminuer de façon directe ou indirecte, la couverture de protection d'assurer, alors même qu'aucune mesure forte dans ce PLFSS permettant un accès effectif. S'il faut soin et un médecin traitant n'est proposée par ailleurs sans solution structurelle pour améliorer de manière globale, l'accès aux soins, les dispositions de l'article 43 ne pourront qu'accentuer les inégalités d'accès aux soins pour des populations peut être les plus précaires ou des populations qui présentent une sur-morbidité cet amendement se propose de maintenir le remboursement des arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une telle consultation via son médecin traitant ou pas dans le cas où le patient résine dans une zone sous-dense, bon, on a un petit échantillon de 110000 pour l'instant, il y a pas vraiment sur le plan statistique d'écart entre zones Soudan ces zones suffisamment doté, moi je les appelle comme ça,

44 % des médecins refusent déjà de nouveaux patients et la situation est particulièrement dégradée dans certains territoires comme l'Allier La Charente, la Seine et Marne, mais il doit y en avoir d'autres, de façon générale, 71 % des médecins interrogés jugent déjà avoir trop de hôtel donc en conséquence il est injuste de pénaliser des populations qui, du fait de leur situation patiente pardon avoir trop de patients, j'aurais dû dire ça comme ça, patiente, il est injuste de pénaliser des populations qui, du fait d'une situation par particulièrement tendue sur le plan géographique peuvent être conduites à recourir à ce dispositif, sans pour autant avoir eu un médecin traitant qui est disponible sur leur zone. Merci. Madame la Sarah le 498. Merci monsieur le président, le principe d'une délivrance d'un arrêt de travail bien sûr en téléconsultation limité au médecin traitant doit être la règle toutefois, il convient également de ne pas pénaliser les patients fragilisés qui sont éloignés des soins cet amendement propose d'autoriser la délivrance d'arrêt de travail en téléconsultation avec un médecin, autre que le médecin traitant dans l'une des conditions restrictives suivantes pour les patients qui vivent en zone sous-dense pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant pour les patients dont le médecin traitant n'est pas disponible dans un délai compatible avec le délai de transmission de l'arrêt maladie. Merci. Madame Sollogoub, le 151. des gens qui ne peuvent pas avoir un médecin traitant qui sont en situation, alors soit ils renoncent aux soins, soit ils ont quand même besoin d'un arrêt mal disons un seul recours c'est celui-ci et qu'on leur dise qu'en plus, ils vont pas être remboursé mais ça va mettre en ce moment ça va mettre le feu aux poudres parce que l'accès aux soins, c'est vraiment le sujet dans les territoires sous-dotés, moi ça va être vraiment très difficile à faire passer, il faut vraiment prévoit alors moi je, je, proposé que, en effet, pour les patients en zones sous-dotées, qui n'ont pas de médecin traitant, il puisse être exonérée de de cette disposition, sinon ça va vraiment, vraiment créer une grosse colère. Merci, avis de la commission sur les trois amendements. prescrit en en téléconsultation des indemnités journalières seraient ainsi bien verser soit l'absence de médecins traitants, soit pour les patients vivant en zones sous-denses, soit les 2 ou enfin si le prescripteur exerce en structures d'exercice coordonné, j'ai pu l'évoquer en commission les difficultés liées aux ondes Soudan sous le soutien aux structures d'exercice coordonné ne sont pas justifiées de permettent des des prises en charge à ce point facilité pour les arrêts de travail, l'équilibre trouvé par cet article et les amendements de commission. Semble le bon à nouveau les consultation du médecin traitant ou d'un médecin vu depuis un an, conserve la prise en charge et tout, mais de sa vie en présentiel bien sûr pourra délivrer un arrêt de travail dans les lui donnant lieu à aux indemnités journalières il faudrait pas que si ces amendements étaient été voté ça pousse certains patients à ne plus déclaré de médecin traitant sous prétexte que ils ont oui mais

Je retire mon amendement, monsieur le président. Vous n'attendait même pas l'avis du gouvernement, votre bien, allez-y, Madame la Ministre, donc il en reste que deux. Monsieur le président, donc un avis défavorable aux deux amendements restant pour 2 raisons, donc la première raison, c'est que l'article n'interdit pas l'indemnisation de tous les arrêts délivrés en téléconsultation je crois qu'il faut être très clair sur ce sujet que l'assuré résidant dans un désert médical pour être indemnisé à la condition de consulter un médecin qui a une connaissance de son dossier médical, nous le maintenons, c'est la garantie d'un suivi médical sérieux, je le répète, un arrêt de travail n'est pas un acte un acte anodin auquel chaque patient va à pouvoir prétendre, quel que soit son lieu de vie, enfin la 2ème raison c'est que le constat de l'assurance maladie et que les patients qui télé consulte ont le même profil que la population générale, ce qui ne manque pas une utilisation plus important de la téléconsultation pour des raisons liées à la disponibilité moindre des médecins traitants dans les zones sous-denses pour ces 2 raisons, un avis défavorable aux deux amendements restant, monsieur le président. Merci Monsieur monsieur le président, je voulais en quelques mots expliquer quelle était notre position, cette question n'a pas déposé d'amendement sur cet article, pourquoi, parce qu'on est tous, je pense à la recherche d'un équilibre entre deux fait de mieux réglementer la téléconsultation qui est actuellement l'objet de dérives et de dérives qui sont significatives mais sans porter atteinte au fait qu'il y a des personnes qui actuellement ne peuvent pas avoir un professionnel de santé, et voilà, si on leur ferme complètement le robinet de la téléconsultation elles ne pourront plus accéder à certaines prestations, donc cet équilibre il n'est pas simple à trouver, le gouvernement a fait une proposition qui est plutôt, on va dire qu'il convient dans l'ensemble, l'amendement 109 de Corinne Imbert et bienvenue pour pour confirmer ce cadrage mais moi je voudrais dire que la téléconsultation c'est devenu un outil de la pratique de soins et donc, il serait sans doute bon de l'intégrer dans la réflexion sur les parcours de soins et pour être encore plus précis que les ministres concernés travaillent avec les organisations de professionnels de santé, les fédérations de patients. Ah élaborer à mettre cette question de la télé consultation comme celle de la PDVSA et discuter, qui est responsable de la PDSA qui l'organise, qui participent, hé ben la télé consultation devrait être une forme de service public de proximité, d'accès aux soins et là où il y a une c'est Pts là c'est BTS pourrait en charge l'organiser, bah, une permanence de téléconsultation pour des personnes qui ne peuvent pas avoir accès parce que elle a raison, Katia pour se polis ou Nadia Sollogoub de dire que c'est un un vrai problème, donc je pense qu'il faut qu'on rentre la téléconsultation dans la chaîne d'organisation de nos parcours de soin, mais ça n'est pas en détruisant les parcours de soins qu'on réglera le problème de la pénurie. Merci. Je vais donc mettre aux voix le 946 2 avis défavorables qui est pour.

l'amendement 100 neuf propose d'encadrer davantage les arrêts de travail prescrits entre des consultations, il vise à prévoir une durée limite pour un arrêt de travail prescrit en téléconsultation et il prévoit également de limiter le renouvellement d'un arrêt de travail prescrit en téléconsultation une nouvelle prescription à l'occasion d'une consultation physique et puis l'amendement 110 hé bien vous propose, madame la ministre d'avancer, d'entrée en vigueur de ce dispositif en mars 2023 je rajouterai pour rebondir. Sur les propos de notre collègue Bernard Jomier c'est que quand tu nous avons discuté de l'article concernant la télé consultation dans les amendements que j'ai proposé, j'ai proposé cette alternance possible entre téléconsultation et consultations en présentiel dans l'idée effectivement d'un parcours de soins qui intègre la téléconsultation c'était un peu de cet esprit là bien sûr ne pas complètement fermer la télé consultation ça n'aurait pas de sens, mais mieux l'encadrer avec une rencontre avec un médecin en en présence physique, ça me paraît quand même la moindre des choses, je vous remercie. Avis du gouvernement sur ces deux amendements 100 910. Alors Monsieur le Président Madame la rapporteure sur le sang neuf un avis défavorable, parce que si nous adoptions cet amendement s'seuls les arrêts de courte durée, donna lieu à indemnisation, ce que vous ne souhaitez pas, je pense que vous souhaitez nous ne souhaitait pas limiter l'indemnisation de tous les arrêts délivrés en téléconsultation, donc, qu'on dirait votre amendement à limiter le droit à prescription des médecins traitants et ce sans justification médicale, c'est pour ça que nous émettons un avis défavorable sur le 110 nous émettons un avis défavorable, mais l'idée est bien d'aller le plus vite possible dans l'exercice de de l'application et de l'encadrement de téléconsultations si nous acceptions votre amendement et si jamais au mois de mars, les services techniques n'était pas en mesure de pouvoir mettre en oeuvre cette c'est cette application, vous nous le reprochent donc qui peut le plus peut le moins, nous avons décidé d'aller jusqu'au mois de juin si les services sont prêts à le faire plus tôt, ils le feront bien plutôt. Merci. Je vais donc mettre aux voix, d'abord le sang 9 de la Commission, avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Qui est contre, il est adopté, je mais voit l'article 46 bisquer pour. Qui est contre, il est adopté. à l'article 47 2 amendements identiques de suppression qui le défend Madame salade. Merci monsieur le président, à l'issue d'un contrôle sur le non respect des règles de facturation, l'article 44 propose de permettre une extrapolation à partir des indus constatés car les organismes de Sécurité sociale ne dispose pas de moyens pour contrôler l'ensemble de l'activité en cause ce transfert de responsabilité est inacceptable et semble aller à l'encontre de plusieurs principes du droit, la disposition semble d'abord aller à l'encontre des droits de la défense, cela revient à renverser la charge de la preuve on imposant à l'administré d'apporter les preuves du respect des règles de facturation, dossier par dossier, sur l'ensemble de son activité de plus, la disposition semble encore aller à l'encontre du droit à l'erreur, instituée par la loi d'une la loi numéro 2008 2018 727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ces articles précise que la preuve de la mauvaise foi, appartient à l'administration, il convient donc de supprimer l'article quarante-quatre. Merci Merci monsieur le président, l'article 44 du PLFSS donc créé de facto une nouvelle peu procédure de sanction des professionnels de santé, à la suite d'un contrôle d'une liste d'activités qui vient s'ajouter aux 5 procédures de sanctions déjà en vigueur pour rappel, l'assurance maladie disposent de la répétition de l'Hindu fondé sur une preuve ressortissants de l'analyse d'activité, la plainte disciplinaire auprès de la chambre disciplinaire la plein disciplinaire auprès de la section de l'assurance maladie, la plainte pénale il y a plein de financière, ces procédures ont été progressivement ajouté pour combattre les fraudes et sont largement à notre avis suffisante à condition qu'elle souhaite appliquer les la disposition projeté donc viendra s'intégrer à l'article L 133 IV du code de sécurité sociale, modifiant substantiellement son application et donnant lieu à 2 alternatives sans que l'on sache quelle modification permettrait à l'assurance maladie de choisir entre 2 procédures, l'Hindu suivant preuve tangible ou par extrapolation, par ailleurs, le texte paraît entre telle contradiction avec l'article L 100 315 tirer hein du grand 4 du code de la sécurité sociale, en pratique, il y a contradiction entre extrapolation et procédure contradictoire quand on extrapole, on soustrait une partie des conclusions à la preuve objective tangible qui permet l'échange contradictoire, il n'est pas certain qu'en soustrayant une partie de l'analyse d'activité au débat contradictoire, la question des caisses d'assurance-maladie soit facilité, bien au contraire, les recours juridictionnel augmenteront nettement dès lors que le praticien mis en cause se verra reprocher des griefs théorique auquel on aboutira pas raccourci celui-là serait progression s'il y a un réel besoin de lutter contre la fraude, il n'y a aucune nécessité, selon-nous d'ajouter une 6ème, procédure qui sera de plus perçu comme culpabilisant merci monsieur le président. Merci. Le 551 n'est pas défendu le 577 monsieur Fiole R. Oui identique : écoutez, moi je n'aurais pas souhaité qu'on corrige mes copies, en prenant qu'un seul exercice sur l'ensemble et qu'on extrapole, s'il était raté à une note globale,

Non, vous n'êtes pas signataire n'c'est dommage pour vous, sûrement, mais vous n'êtes pas signataire le 851 madame Jacques, il est défendu, merci le 948 madame poncer Monge. Oui, alors il reste plus grand chose, j'essaie de voir 2 complémentaire à dire sur cette demande de de suppression, mais effectivement moi je pour conclure enfin la disposition sommes quand même aller à l'encontre des droits de l'établissement, mise en cause, alors on a dit ça revient renverser la charge de la preuve mais même après recours en fin de compte, l'établissement n'auraient, comme seule solution : l'établissement de santé d'apporter les preuves du respect des règles de facturation, dossier par dossier, donc ça c'est, c'est c'est lui qui. Sera le le travail un petit peu exhaustif pour prouver sa bonne foi, sur l'ensemble de son activité, donc bon, que dire de plus, enfin bon, moi, je pense aussi qu'il y a un contexte aussi a proposé, dans un contexte quand même, on connaît les l'état de nos établissements de santé, de faire peser une pression accrue sur la question du codage ou quelques fois il y a des quand même de réels problèmes d'interprétation, alors vous allez me dire ça, c'est le contradictoire avec la menace de sanctions financières bien supérieures à celles connues à l'heure actuelle, parce que quand même l'objectif je pense c'est d'augmenter les sanctions financières alors que même que les établissements s'interrogent sur leur soutenabilité financière bon outre d'État un dispositif là ça a été largement développé pas recevable il fragilise de plus, la situation des hôpitaux notamment. Merci.

monsieur le rapporteur sur ces amendements identiques. Quand nous avions examiné cet cet article et au niveau de la commission, nous étions dans la stratégie que nous avons continué

de. Six sien ou bien d'établissement, c'est la raison pour laquelle nous avons donné un avis favorable. Mais nous avons bien compris que

Concernés par ces indus, merci, je vais essayer de vous donner les motivations de, de, de la commission par rapport à cela puisque cet amendement vise à supprimer donc cet article qui permet aux directeurs de CPAM de fixer forfaitairement le montant d'un indu par extrapolation des résultats du contrôle d'un échantillon de de facture très bien alors je voulais vous dire ici que la procédure prévue, que nous avons examiné quand même de près hein pour répondre en partie à vos questions, la procédure prévue pour le recours à cette faculté est particulièrement encadrée et nous a-t-il semblé garantit les droits de la personne contrôlée, il s'agira avant tout de repérer une méconnaissance régulière des règles de facturation de distribution ou de tarification ainsi la fixation forfaitaire du montant de l'Hindu ne pourra intervenir qu'au terme d'une procédure contradictoire avec le professionnel, le distributeur ou l'établissement concerné au surplus la somme fixée au terme de cette procédure ne sera opposable aux 2 parties que lorsque son montant montant aura été validé par écrit par le professionnel, le distributeur ou l'établissement dans le cas contraire, une procédure contentieuse pourraient être engagée dans le but de contester ce montant. Nous pensons nécessaire de donner aux agents des organismes de Sécurité sociale, tous les moyens une disposition pour leur permettre d'accomplir dans les meilleures conditions leur mission et en particulier de lutte contre la fraude, en effet, la fraude sociale porte une atteinte intolérable au principe de solidarité et affaiblit considérablement le consentement de nos concitoyens au paiement des cotisations sociales, c'est la raison pour laquelle il nous semble important d'agir pour que ces comportements. Module cesse voilà il y a quand même une concertation, une discussion, ça en fait, me semble-t-il, me semble-t-il, donner un rôle de médiateur un peu aux directeurs de CPAM pour quand y a constatation d'un du répétés sur des fraudes bien bien que il y ait cette discussion qui permettent que les caisses de Sécurité sociale puisse retrouver l'argent qui aurait été. Indûment détournés, alors je me tourne vers le gouvernement, hein : comment une mesure qui semble techniquement tout à fait pertinente peut être mal vécue par l'ensemble des professionnels des établissements qui ont vraiment le sentiment de d'être soupçonné, a priori, et même de de fraude, nous les avions auditionnées effectivement ils étaient quand même unanimement pour nous demander de prendre d'autres mesures, mais en tout cas jugé celle-là, celle-là tout spécifiquement particulièrement. Désagréable vis-à-vis des de leur profession ou de leur établissement, donc nous attendons vos explications non, Monsieur le Ministre. Attendez monsieur l'emportèrent là parce que d'un côté, vous dites que voilà et ensuite vous interpeller en fait qu'elle est la vie, alors c'est une bonne question. Monsieur le président je pensais y échapper mais la vie, la vie bon l'avis de la commission est défavorable et je me suis permis d'attirer l'attention du gouvernement

Merci monsieur le président je pense que c'est important qu'on s'arrête un instant sur effectivement cet article puisque je vois que la quasi- totalité des groupes de cet hémicycle ont déposé des amendements de suppression, je pense que ça fait écho par ailleurs effectivement à des inquiétudes qui ont été relayées par certaines fédérations hospitalières ou de professionnels de santé, et moi je vais essayer de vous convaincre, je suis pas sûr d'y arriver mais je pense que c'est important. Ton monde essayer puisque je ne peux pas croire que dans cette haute assemblée qui a fixé la lutte contre la fraude, les abus et les indus comme une grande priorité avec l'adoption d'une proposition de loi que j'évoquais tout à l'heure qui a quand même régulièrement suivi aussi les rapports de la Cour des comptes sur ce sujet-là, qui est par ailleurs extrêmement attentive à la bonne gestion des finances publiques et à ce que les deniers publics soient utilisées de manière la plus efficace possible, je ne peux pas croire que, il y a une opposition de principe à cet article qui permet une meilleure gestion de l'argent public c'est exactement de ça qu'on parle en coordination avec des propositions qui sont faites par la Cour des comptes et en coordination aussi avec un principe qui a été introduit dans le droit de la sécurité sociale par le PLFSS de 2016, à l'époque où le gouvernement était socialiste et donc je pense que, lutte contre la fraude de l'ensemble des fraudes des indus par ailleurs des mesures qui ont été portées dans un autre quinquennat cela deux pourrait vous faire vous retrouver autour de ce sujet là de quoi on parle, on parle du contrôle des factures payées par l'assurance-maladie est ce qu'on pense que l'assurance maladie est capable de regarder une à une, l'ensemble des factures qui sont délivrés pour l'ensemble des professionnels de santé pour l'ensemble des établissements de santé, évidemment non, et ça on le sait tous, il y a une atomisation absolue des factures selon les axes, selon le type de séjour et vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers de facture aujourd'hui l'assurance maladie, elle a le droit d'extrapoler, donc elle a le droit de contrôler sur un échantillon de factures et de regarder s'il y a des indus, exemple, un acte qui serait mal côté et qui aurait entraîné de l'argent public qui auraient été un établissement ou un professionnel de manière de manière indue aujourd'hui l'assurance maladie ne peut récupérer ce qui est étendu que sur la période concernée par l'échantillon de facture, or on sait bien que sur un certain nombre de cas, c'est parfois même une erreur hein je j'en conviens, totalement, mais une erreur de cotation qui n'est pas limité à l'échantillon temporel des factures qui sont contrôlés, mais qui a qui qui qui qui existe depuis plus longtemps et donc ce que cet article prévoit, c'est de donner la possibilité aux caisses d'assurance maladie de demander le remboursement de l'Hindu sur une période qui va au-delà de l'échantillon qui a été regardé quand on sait qu'on a matériellement la possibilité de savoir que c'est un un du qui a cours depuis plus longtemps, ça ne dit ni plus ni moins que ça, et je pense que chacun peut le comprendre, on ne parle pas par ailleurs de sanction de punitifs on parle là de gestion des ennuis, c'est une mesure de gestion plus qu'une mesure de lutte contre la fraude, d'ailleurs, mais quand il y a de l'argent public qui est versé indûment que c'est matériellement attestée par un contrôle de l'assurance maladie et bah, si ça me paraît légitime que l'assurance maladie puisse demander à récupérer l'ensemble des sommes qui ont été versés indûment ce que prévoit cet article, je pense que là où il y a une inquiétude des fédérations et de certains professionnels, c'est sur l'absence de respect du contradictoire, ça a été relevée par un certain nombre d'entre vous en gros que l'assurance maladie arrive et dise on a détecté sur notre échantillon de facture sur telle période qui avait tel on on imagine que bah c'est un un du qui existe depuis plusieurs années, donc on va vous demander de rembourser davantage et que l'établissement n'est pas la possibilité de répondre, évidemment qu'on prévoit pas ça du tout, évidemment qu'il y aura une procédure qui a une procédure prévue de contradictoire avec l'établissement en question et je pousserai même plus loin en disant que si l'établissement en question n'est pas d'accord avec le remboursement d'un du qui lui est demandé par l'assurance maladie, il a tout à fait la possibilité de saisir la justice pour contester le montant qui lui est demandé ce qui simplifierait pas la la vie de l'administration pour vous répondre les c'est le non mais pour vous répondre Monsieur Bruillet ce qui ne simplifierait pas la vie de l'administration, c'est si on considérait que l'administration de regarder chacune des centaines de milliers de factures qui sont aujourd'hui réalisés pour des professionnels ou des établissements de santé, je me souviens que la semaine dernière j'étais dans cet hémicycle, il y a un amendement qui a été adoptée pour supprimer des postes de fonctionnaires alors moi je veux bien qu'on recrute des milliers ou des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires pour contrôler chaque facture qui est versée par l'assurance maladie à chaque professionnel de santé et chaque établissement de santé, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on serait dans la bonne gestion des deniers publics, donc c'est un article de bonne gestion et et, croyez bien et toutes les garanties, puisqu'on l'a aussi échangé avec elle et continueront à donner sur le respect du contradictoire, il s'agit pas, on a encore une fois dans le punitifs, il s'agit juste de permettre à nos finances publiques, de récupérer des sommes indues, encore une fois, à un moment où chaque Euro compte donc j'espère sincèrement que ces amendements pourront être et que l'Arctique pourrait être voté. Vous avez le droit d'espérer Monsieur le Ministre, alors j'ai Monsieur Jomier plus Madame Prima, mais si tout le monde va dans le même sens, on va peut-être pas faire prolonger le débat,

vous avez raison, monsieur ministre de rappeler que ça existe déjà dans notre droit et vous, vous vous n'introduisait pas un principe nouveau avec l'extrapolation seulement ce type de principe enfin ce type de de de méthode doit être très strictement encadrée parce que elle est pas exorbitant du droit commun et je voudrais pas employer des mots trop forts, mais quand même dérangeante au regard du droit commun, or d'exposer de René-Paul Savary est très très illustratif, ça a été très compliqué pour lui, nous expliquer que tout ça était très bien cadré et en fait ça ne l'est pas très bien cadré et introduire, alors quel est l'intérêt d'introduire d'étendre ce Champ de l'extrapolation si ça allait pas très bien cadré, on le lit dans l'étude d'impact, hein, et vous en avez, vous avez un peu abordé le sujet, pour des raisons de RH, c'est-à-dire bon bah, ça fera moins de personnel, ou autrement dit, avec le même nombre de personnels on contrôlera plus

autour de quelques millions d'euros, c'est pas négligeable, quelques millions d'euros, mais moi je dis nous, nous disons que le jeu n'en vaut pas la chandelle que et étendent le Champ de l'extrapolation de façon si mal cadré pour récupérer quelques millions d'euros pour une année sur tout le territoire national, non, il vaut mieux revenir l'année prochaine avec une proposition mieux mieux établie. Merci monsieur le Président, je vais essayer d'être rapide, alors comme je ne suis pas une grande spécialiste du PLFSS j'ai reregardé le texte et quand je lis l'inobservation des règles et lorsque l'inobservation des règles et révélé par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel est fixé faut forfaitairement par extrapolation tout ou partie de l'activité d'lieu à la prise en charge de l'assurance maladie et caetera, il me semble qu'en effet, les propos de monsieur sont justes, c'est pas très très cadré, moi je suis pas sûr de comprendre exactement si le professionnel à qui on va redemander des indus et vous avez raison, il faut le faire, parce que si il y a eu une erreur ou s'il y a eu une difficulté, il faut, il faut évidemment l'État retrouve ses ses petits mais je trouve que forfaitairement par extrapolation, ça permet pas un cadrage dans la durée, dans la profondeur, ça on comprend pas bien de quoi il s'agit donc moi je, je ne sais pas, mais on ne sait pas terminé le PLFSS là il va y avoir quand même des discussions après donc, peut-être qu'on peut mieux encadrer cette disposition là pour rassurer les professionnels qui semble pas du tout rassuré parce que si on partage le même amendement partout, c'est qu'il y a probablement un problème donc il me semble que dans la suite de nos travaux, on peut être un peu rassuré les sénateurs et les parlementaires d'une façon générale, et les professionnels surtout. Monsieur le rapporteur. Oui merci l'extrapolation, on l'a dit existe déjà, on l'applique, par exemple quand il y a la constatation d'un indu envers un professionnel ou un établissement pour les pénalités vous avez un indu de temps on dit probablement c'est prenant l'erreur de cotation, puisqu'elle avait pris par Monsieur le Ministre, ça s'applique depuis 2 3 ans, et donc en conséquence, vous aurez une et pénalités qu'on va calculer en en fonction de l'extrapolation n'pas la récupération de l'Hindu

Il y a une manière de faire. Voilà une manière de faire et on vient pas me semble-t-il, comme ça, envoyer un professionnel une lettre en disant : voilà, on a constaté des indus on extrapole toc et vous nous devez étant après lance une discussion. Parce qu'il y a discussion, mais simplement on peut peut être les alerter qu'on a constaté quelque chose et qu'on rentre en discussion pour leur dire : voilà ce que voilà, la façon dont on fait je veux dire, oui c'est prévu sauf que si il y a 7 c'est, c'est cet esprit de suspicion et quand on, quand on interroge des professionnels, hein, puisque ça existe déjà, l'extrapolation qu'ont été soumis justement à ce contrôle et ben on arrive en disant : voilà, vous avez fraudé, c'est la raison pour laquelle je pense que il y a une manière de faire pour arriver à ce qu'il y ait pas ce sentiment de suspicion, c'est comme ça qu'on arrivera parce que c'est pas le tout de voter la loi, si elle est pas appliquée,

allez, et puis merci, monsieur le rapporteur, mais enfin, vous donnez un avis défavorable aux amendements et après vous les expliquez moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est pas simple pour ensuite provoqué le vote, monsieur le ministre, une dernière intervention je mets aux voix les dix amendements identiques. moi c'est pour répondre aux aux interventions qui ont eu lieu, encore une fois aujourd'hui le droit nous permet de faire une extrapolation le droit permet aujourd'hui à l'assurance maladie de demander à un échantillon de facture sur une période donnée, et lorsqu'on constate un un du, par exemple, un acte qui est mal codé de récupérer les indus sur cette période, ça, c'est ce qui existe ce qu'on dit, c'est que dans un certain nombre de cas, on voit que les actes sont mal codé depuis plus longtemps que ceux-là, c'est quelque chose de répétitive et donc on donne la possibilité, via cette extrapolation de récupérer des indus antérieures à la période d'échantillonnage des factures et ça se fait, pour le coup, de manière totalement encadrée par le droit de presque de prescriptions qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire 3 ans s'il s'agit d'un du je crois 5 ans s'il s'agit de fraude, mais encore une fois, moi, je veux dire que il s'agit pas de dire que l'assurance maladie va arriver, il va dire vous nous devez tant

à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance-maladie et ce professionnel ce distributeur ou cet établissement, donc le fait qu'il y aura une procédure contradictoire il y figure dans le texte même de cet article, ce qui pour moi est de nature à rassurer quand même sur le fait qu'il sera évidemment respecter encore une fois, il s'agit simplement de bonne gestion de l'argent public, moi j'entends les inquiétudes sur la stigmatisation général quand ces arguments là sont manier pour d'autres types de fraudes ont dit il ne faut pas à vous, enfin voilà ça peut pas être un argument pour ne pas agir, et cetera, je pense que voilà, il ne faut pas non plus que ce soit un argument qui nous pousse à ne pas donner des leviers pour récupérer de l'argent public qui a été versé indûment Merci. Bien, je vais mettre aux voix, donc les 7 amendements identiques de suppression de l'article, qui reste avec un avis défavorable du gouvernement et un avis défavorable de la commission, même si bon, allez, qui est pour ces amendements de suppression. suppression. Ces amendements sont adoptés, l'article 44 et donc supprimer fait tomber naturellement les cinq amendements qui suivaient sur l'article.

Merci monsieur le président, le présent amendement a pour objet d'apporter une contribution positive au débat en prévoyant parallélisme des formes avec le même cas de figure pour les professionnels de santé libéraux que la commission de contrôle compétente pour avis soit constituée à parité de représentants des financeurs, d'une part et de représentants des fédérations hospitalières publiques et privées, d'autre part, telle est en effet le cas pour la Commission au de l'Arctique L 162 1 14 du code de la Sécurité sociale qui prévoit, dans sa deuxième phrase, lorsque, lorsque est en cause, une des personnes mentionnées au 3ème alinéa du hein, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission, il faut mesurer la complexité des classifications et de leurs règles de codage pour comprendre les limites de certaines interprétations et le désarroi ou le sentiment d'injustice devant la définition de certains qualifié, qualifié, quelquefois de fraude et le poids des sanctions parfois infligés de manière disproportionnée, le rééquilibrage logique de la commission de contrôle permettrait d'établir un cadre commun et utile de discussions des situations assurant une meilleure évolutivité et acceptabilité du dispositif en conclusion à la présente proposition d'amendement vise à assurer une composition paritaire des commissions de contrôle de la tarification à l'activité entre représentants des financeurs et des fédérations hospitalières publiques et privées, à l'instar du dispositif existant pour les professionnels de santé libéraux afin de favoriser la compréhension et la diffusion optimale de l'information entre les parties prenantes, tout en garantissant tant la justesse que la légitimité des avis produit.

aux règles de facturation, il s'agit en particulier de prévoir que cette commission est présidée par un magistrat et qui siègent des représentants des fédérations hospitalières représentatives, publics ou privés, la composition actuelle de la commission constituée à parité de représentants de l'ARS et des organes mine d'assurance maladie et du contrôle médical nous semble à la fois cohérentes et représentatives des intérêts en présence, du reste, je rappelle que le directeur de l'aérien et ce n'est pas tenu par l'avis de la commission, en conséquence, nous émettons un avis défavorable.

de demander un rapport au gouvernement sur l'octroi de trimestres complémentaire aux élus locaux, à l'occasion du calcul de leur retraite, lors des élections municipales de nombreuses communes ont connu des difficultés de constitution des listes de candidats et il s'agit d'aligner le dispositif qui a été voté en faveur des responsables associatifs et bénévole à l'initiative du député Yannick Favennec en faveur des élus locaux, je vous remercie. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Effectivement, c'est un sujet important que de prendre en compte effectivement les mandats d'élu mais c'est un rapport et vie donc négatif sujet à avoir au moment de la réforme sur les retraites bien entendu.

Alors. C'est un demande de de rapporte donc l'amendement d'appel, la protection sociale des Français établis hors de France est essentiel en terme de justice par rapport aux autres, aux autres Français, il est impératif de réformer notre système social afin que travailler à l'étranger ne soit plus pénalisant et assure une égalité de traitement rendent celui-ci plus équitable nécessite une refonte du calcul des retraites. Par exemple, en calculant le salaire annuel moyen à partir des meilleures années travailler en France ou en supprimant la décote véritable double peine pour les carrières courtes qui concernent notamment des femmes ayant suivi leur conjoint à l'étranger s'ajoute que l'État participe à financer le dispositif dit de 3ème, catégorie de 3ème catégorie des de la caisse des Français de l'étranger qui vise les personnes aux revenus les plus faibles, mais cette participation est passé de 50 % lors de la création du dispositif en 2002 à environ 10 % aujourd'hui mettent en danger sa pérennité, le faible nombre de bénéficiaires du dispositif est également inquiétant et pose question sur l'accessibilité à ce dispositif, alors que le dernier rapport du gouvernement 2020 sur la situation des français établis à l'étranger, rapporte une précarisation croissante réfléchir à supprimer le seuil minimum de 15 ans de cotisation pour prendre en charge tous les retraités français résidant à l'étranger, garantir l'accès à la caisse des Français de l'étranger pour les foyers les plus modestes ou encore pérenniser les aides sociales exceptionnelles des consulats dans un véritable fonds de solidarité nationale, sont autant de pistes pour que la solidarité nationale soit étendue à l'ensemble des situations parfois douloureuses auxquelles sont confrontés les Français vivant à l'étranger, c'est pourquoi le présent amendement vise à présenter au Parlement un rapport sur les améliorations à apporter la protection sociale des françaises et tu as des Français et Françaises établis hors de France, et là je trouve vraiment très utile, un rapport vu quand même l'évolution très préoccupante de la situation des Français établis hors de France, avis de la commission. Oui, merci d'avoir soulevé ce problème qui est particulièrement important et qu'il faudra surtout aborder au moment de la réforme des retraites, donc avis bien sûr défavorable sur la demande de rapport, malgré l'intérêt du sujet. Avis du gouvernement, même avis pour les mêmes raisons merci dans 66 avec 2 avec 2 avis défavorables. Qui est pour.

Pardon, monsieur le président, chers collègues Monsieur le mini-chers collègues, ma collègue Mélanie Vogel a eu l'occasion de le dire, l'intégralité des amendements de notre groupe vise à construire une sécurité sociale, écologique, c'est-à-dire un modèle de protection sociale adaptée au risque d'aujourd'hui qui pèse sur notre santé, nos parcours professionnel et nos vies. Ils aggraveraient la dépense publique, alors qu'à l'inverse, la prévention s'auto-finance largement à moyen terme, cette vision étriquée nous pousse adopter des textes inadaptés face aux grands défis du siècle, la crise climatique et environnemental, ne pas mettre en place des mesures préventives aggraverait non seulement la dépense publique, mais aussi l'état de santé de la population et notre qualité de vie, les crises à venir, par leur ampleur et leurs coûts sociaux et humains peuvent mettre en danger des acquis sociaux, si notre système de santé ne s'adapte pas les risques environnementaux sont aussi des risques sociaux qui touche avant tout les plus vulnérables, ils ne vont que s'aggraver si nos politiques publiques ne change pas radicalement pour faire face à ces enjeux et ses bouleversements, le Sénat a adopté en avril dernier un rapport sur la mise en place d'une sécurité sociale, écologique, c'est dans cette perspective et parce que les propositions concrètes qui existe n'ont pu être débattu pour cause d'irrecevabilité que cet amendement a été déposé, il demande un rapport au gouvernement pour évaluer les pistes permettant de maintenir la sécurité sociale comme pilier de la protection de nos concitoyens et la redistribution comme levier majeur de compensation des effets de certaines politiques de transformation écologique pour en accélérer l'acceptabilité et atténuer les effets, c'est donc une demande de rapport. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Avis défavorable puisqu'il y a à la question et la réponse à l'intérieur de l'amendement, il y a un rapport qui a été publié, c'est pas la peine d'en faire, oui du gouvernement. Oui, mais ma vie et j'avoue et j'ajouterai, parce que c'est mentionné dans l'exposé de cet amendement, que la question de la prévention est absolument central et majeur, et tout l'enjeu de ce qu'on cherche à construire, c'est évidemment faire évoluer nos politiques de santé, la sécurité sociale pour prévenir plutôt que guérir davantage dans la prévention que dans le curatif, vous aurez noté que la prévention figure désormais dans le titre des attributions du ministre de la Santé, qui est ministre de la Santé et de la prévention et évidemment, ça se traduit aussi dans toutes les politiques on impulse notamment dans ce PLFSS. Merci le 967 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre rejeté. Article 45 madame la rapporteure, un amendement de la commission cent merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour objet d'une part, de fixer le principe de la fixation par la loi, c'est-à-dire en pratique par la loi de financement de la Sécurité sociale, du montant des dotations de la sécurité sociale en 1er lieu de l'assurance maladie à l'ensemble des fonds et organismes qu'elle subventionne les demandes devront ainsi être au premier euros devant le Parlement, je vous le rejoint, Monsieur le Ministre, hein, chaque Euro compte, il s'agit d'un principe de base de bonne gestion des finances publiques dont l'application de longue date pour les finances de l'État n'empêche pas le bon fonctionnement dans quel opérateur dans la rédaction proposée tout texte législatif par exemple une loi d'urgence pourrait servir à rectifier le montant de la dotation en cours d'exercice, si cela se révélait nécessaire même si le dépôt d'un collectif social serait bien sûr la meilleure manière de procéder, d'autre part, cet amendement propose d'octroyer formellement cette dotation pour Santé publique France alors que l'agence fait l'objet depuis 2020 de dotation exceptionnelle de plusieurs milliards d'euros par an des voyant le principe d'autorisation parlementaire de la dépense et sans qu'il en soit rendu compte aux commissions chargées de l'examen des lois de financement, il est ménagé une dotation exceptionnelle correspondant à la provision inscrite dans l'à 2023. commission. Ce président madame la rapporteure, comme vous le savez, dans un souci d'une meilleure information de la représentation nationale les annexes de la FSS ont été enrichi afin de présenter les dotations accordées par l'assurance maladie aux opérateurs de l'État pour l'année à venir, en plus de l'année en cours et de l'année passée, l'annexe 2 du présent Plfss comporte déjà et c'est la première fois les informations relatives à la dotation des opérateurs financée notamment par le sixième sous l'objectif de l'Ondam, vous le savez, cette nouveauté récente est issu de la loi organique du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la Sécurité sociale et nous ne souhaitons pas revenir sur l'équilibre qui avait été trouvé à cette occasion concernant santé publique France le fait de pouvoir financer ses moyens on par arrêté, a permis de réagir, notamment pendant la crise sanitaire et d'aller au plus proche des besoins de de cette de santé publique France donc nous émettons un avis défavorable à votre amendement. Merci. Madame la rapporteure générale. permis de faire de premiers progrès l'annexe de nous informe désormais des lignes budgétaires pour 2023, ce qui est bien le moins au moment où nous votons les objectifs de dépenses pour 2023 mais semblait inconcevable il y a encore un an, je vous le rappelle, de plus, nous serions immédiatement informé en cas de dépassement de ces enveloppes de plus de 10 vu d'où nous venons, ce Vert aux cars pleins vaut mieux qu'un verre vide mais il convient de renforcer encore le contrôle du Parlement sur ces crédits, singulièrement pour ce qui concerne Santé publique France nous entendrons prochainement la Cour des comptes à qui notre commission a demandé un rapport sur cette agence sans vouloir tirer de conclusions hâtives avant cette audition, une évidence s'impose dans ces domaines de compétence, l'agence est le bras armé de l'État, la tutelle est exercée par le seul ministre chargé de la santé et la direction générale de la Santé l'assure au quotidien, bref les ça l'État décide de tout, et la sécurité sociale ne décide de rien, or s'agissant du financement de santé publique, France, la sécurité sociale paye tout et l'État ne paye plus rien depuis 2020, cette différence décideurs payeur étant soit profondément anormal, mais il est encore plus anormal que le gouvernement en profite pour s'exonérer de ce qu'il aurait dû faire, si l'État avait conservé la responsabilité du financement de santé publique France revenir devant le Parlement, quand il est nécessaire de réclamer une rallonge de plusieurs milliards d'euros, plusieurs années de suite surtout quand une partie non négligeable de ses crédits est ensuite reversée à l'État lui-même au travers de fonds de concours, ce qui constitue un véritable dévoiement du principe d'autorisations budgétaires cet amendement et donc un rappel des plus élémentaires pratique de bonne gestion, qui ne doivent pas disparaître comme par enchantement dès lors que c'est la sécurité sociale qui paye, j'y insiste, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, j'invite donc l'ensemble du Sénat à le soutenir. Hé bien je mais on voit le 113, donc de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il est adopté, je mets aux voix, l'article 45 est pour. Qui est contre.

au fonds de modernisation pour l'investissement santé destiné au refinancement, centres de santé, pourquoi, parce que le refinancement descendent de santé se justifie, compte tenu des risques très importants de fermeture et donc de rupture de soins dans les territoires, lesquels sont engendrés par un déséquilibre économique liée à de nombreux facteurs que je ne cite pas, mais qui sont aussi liées à à ce qu'on appelle les trous de la raquette du Ségur de la santé, je vous remercie. Merci. Avis de la commission

au fond de modernisation pour l'investissement santé destiné au refinancement des centres de santé, mes chers collègues, vous le savez, au niveau de notre groupe, nous sommes des ardent des défenseurs des centres de santé convaincu par ce modèle de structure, tant en termes d'accès aux soins que pour les conditions de travail, avec un mode d'exercice en équipe regroupée coordonnées de plus, les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1 sans dépassement d'honoraires et sans avance de frais, reconnue par le code de la santé publique aux articles L. 63 23 tirer hein, ils permettent à la fois un recours à des soins de proximité tout en offrant des soins plus complexe, on a vu notamment le rôle essentiel durant la crise sanitaire, malheureusement pour nous, les Centres de santé sont souvent oubliés ou en tout cas, monsieur le Ministre, Madame la Ministre, pas suffisamment je l'ai évoqué notamment en terme de financement lors de la présentation de la motion du groupe CRCE lundi dernier, la nécessité de refinancer les Centres de santé se justifie par des risques très importants de fermeture et donc de rupture de soins engendrés par un déséquilibre économique liée à plusieurs facteurs, la non-transposition des dispositifs d'aide au Centre de santé à l'identique des mesures d'aides attribuées aux professions professionnels libéraux de la non prise en compte d'un mode de fonctionnement spécifique lié à leur nature même de structures pluridisciplinaires à même de mettre en place un parcours de soins coordonnés trois l'absence de revalorisation financière de leur professionnel de santé pour faire suite aux Ségur de la santé, accroissant leurs difficultés de recrutement et de fidélisation de leur personnel, tous ces éléments donc justifie amplement notre amendement qui j'espère sera votée. Merci. Madame la rapporteure. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 40 de la loi de financement pour 2001 modifié par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 prévoit bien au titre des missions du Fonds pour la modernisation et l'investissement santé le financement des dépenses d'investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire mais aussi des structures d'exercice coordonné les centres de santé étant bien mentionné dans les renvoie au code de la santé publique, cet amendement apparaît ces amendements apparaissent donc satisfait même sur le fond il est occasion c'est d'interroger le ministre sans pouvoir prolonger le débat sur l'utilisation des crédits du mais Potel pourra-t-elle nous nous répondre par écrit, en tout cas, puisqu'ils sont tous les 2, satisfait, c'est une demande de retrait, à défaut, un avis défavorable. Merci madame la ministre. Même avis que la rapporteure. Merci. Je vais donc mettre aux voix, ces 2 amendements identiques avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Rejeté. Je mise aux voix, l'article 49 qui est pour. Qui est contre, Adopté après l'article 46 le 1103 Madame le héros. Merci monsieur le président, il s'agit d'un amendement d'appel hein sur le dispositif MonPsy qui a été introduit par la loi de finances de Sécurité sociale de 2022, et qui prévoit le remboursement d'un nombre limité de consultation d'un psychologue, à condition qu'elle soit prescrite par le médecin traitant ce rapport permettra d'évaluer l'opportunité de supprimer l'adressage par le marché, l'instauration de l'obligation d'une consultation d'un médecin préalable à celle d'un psychologue ne vient aucunement faciliter l'accès aux psychologues, ce qui était pourtant le postulat de départ, c'est au contraire une complexification notamment pour certaines tranches d'âge des 18 35 ans qui est instauré, ainsi qu'un coup, il induit induit inutile l'instauration de cet intermédiaire supplémentaire pour provoquera nécessairement un allongement du délai pour accéder aux soins en psychologie voire empêchent l'accès au dispositif du fait de la pénurie de médecins pour lutter contre la difficulté d'accès aux soins, le choix a été fait à plusieurs reprises d'ouvrir ou d'expérimenter pour des professions de santé prescrite un accès Direct, notamment dans le cadre de la loi de 2000 PLFSS 2022, ces mesures auront terme nécessairement pour effet de libérer du temps médical au profit des patients, suite à l'instauration de cette mesure, à ce jour, ce sont près de 2000 psychologues qui ont intégré ce dispositif sur 15000 professionnels, ce qui est peu, et moins que ce qui était attendu, il convient donc de tracer des pistes d'amélioration : suppression de l'adressage préalable du nombre plafond de séances de psychologue parce qu'il y a aussi un un nombre limité, pris en charge par an du conventionnement préalable avec les professionnels concernés, ainsi que de la fixation d'un, d'une durée plafond des séances, prise en charge, merci. Merci, il avait. La commission. Nous avons à plusieurs reprises lors de nos débats, monsieur le Président évoquer ce dispositif MonPsy notamment quand nous avons discuté, l'article 25 certains amendements demandé sa suppression, d'autres rapports, donc ça reste une demande de rapport en l'état, et c'est toujours un avis défavorable. Avis du gouvernement. la santé mentale de de nos concitoyens sur ce dispositif particulièrement une évaluation est prévue en 2025 et donc votre demande de rapport ben faut laisser un petit peu le temps au dispositif de se mettre en place, il vient de se mettre en place l'idée vraiment de l'évaluer, de laisser s'installer dans le temps de l'évaluer et de de mettre en place la place des psychologues dans la prise en charge de la santé mentale de nos concitoyens, donc je considère que votre à votre demande d'amendement, d'abord c'est un rapport mais surtout est satisfait donc retrait sinon rejet défavorable.

à l'article 46 bis Madame Cohen. qui vivent sous le même toit que des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active mais qui ne sont pas considérés comme étant à leur charge, pour le bénéfice du RSA ne bénéficie actuellement pas de la complémentaire santé solidaire, il s'agit donc d'élargir l'attribution automatique de la complémentaire santé solidaire gratuites mises en place depuis janvier 2022 pour les bénéficiaires du RSA à ces jeunes, ils bénéficieront également du renouvellement automatique de leur droit à 7 complémentaires, de même pour faciliter le recours des bénéficiaires de l'ASPA, l'article 88 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, a mis en place à compter du premier avril 2022 une présomption de droit à la complémentaire santé solidaire participative pour les bénéficiaires, donc de l'ASPA, qui n'exercent pas d'activité professionnelle cette présomption de droit simplifier leurs démarches de demande, il s'agit d'temps de cette présomption aux éventuels conjoint, concubin concubin ou partenaire des bénéficiaires de l'ASPA dès lors qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, ces avancées allant dans le sens d'une meilleure prise en charge des publics fragiles, nous les soutenons. Merci le 114 madame la rapporteure. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est un amendement de clarification rédactionnelle du droit automatique des jeunes majeurs rattachés à foyers allocataires du RSA de bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Le 114 de la commission avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il est adopté, je mais voit l'article 46 bisquer pour. Qui est contre, il est adopté. à l'article 47 2 amendements identiques de suppression de l'article d'abord Madame Cohen. Merci monsieur le président, l'Arctique 47 prévoit l'objectif de dépenses pour l'assurance maladie pour 2023, fixé à 3 7 % soit un niveau inférieur à l'inflation, nous en avons longuement parlé, mais également aux besoins, il manque 1,3 milliards d'euros aux hôpitaux pour tenir compte de l'évolution naturelle des dépenses, la fin de la pandémie signe donc le retour des politiques de compression des dépenses de santé des hôpitaux qui se concrétise et vous le savez, par des suppressions de services des fermetures d'établissements, des suppressions de lits d'hospitalisation, bref une réduction de l'offre de soins hospitalière, c'est ainsi que l'on voit partout des établissements qui craque pour toutes ces raisons et parce que nous en avons longuement parlé, nous demandons la suppression de cet article. Merci 950 Madame. Merci monsieur le président, donc, malgré une augmentation des moyens attribués à l'Ondam, force est de constater que le compte n'y est pas et que notamment le montant de l'Ondam hospitalier sous-évalué l'Inter- fédérations hospitalières estiment que l'inflation n'est prise en compte. Que pour 2 tiers que les surcoûts Covid d'ailleurs, sur la base n'ont pas été totalement compensé ce qui obligera à des économies pour compenser cette sous-estimation invalidant le récit d'un don d'âme sans exigence d'économie, les fédérations unanimes, estime qu'il manque un milliard ça vient d'être dit, ah l'Ondam hospitalier, ce qui implique autant d'économie des établissements dont beaucoup dans le public et le privé non lucratif sont déjà au bord de l'effondrement, la comptabilisation de l'Ondam annuel empêche les établissements hospitaliers de se projeter dans un financement pluriannuel capable de résister aux crises sanitaires potentiels et répondant enfin aux besoins de santé territoire par territoire, la fermeture des maternités de proximité, la transformation des centres hospitaliers ont en hôpitaux de proximité sans maternité chirurgie et urgences, la fermeture de lits d'hospitalisation d'hospitalisation complète la fusion d'hôpitaux, l'introduction de nouvelles formes de management centrée sur la réalisation d'économies résulte d'une logique comptable qui préside et et oriente son dame en rupture avec les aspirations des salariés, un travail de qualité auprès des patients, nous avons besoin d'un choc d'attractivité et donc d'une grande loi de santé appuyé sur une programmation pluriannuelle de financement par cet amendement d'à peine, nous demandons à reconsidérer en profondeur les logiques austéritaires qui ont présidé à l'établissement de l'Ondam, jusqu'à présent et d'un financement des établissements de santé à partir, enfin d'une logique des besoins des territoires de santé. S'il y avait de la commission madame la rapporteure. merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, la commission est défavorable à ces deux amendements de suppression, nous voulons avoir le débat sur l'Ondam, donc voilà, avis défavorable. Avec du gouvernement. madame la sénatrice par rapport à ce que vous avez dit, quand vous avez parlé de politique austéritaire très sincèrement je, je suis ministre du Budget, donc évidemment quand on dépense de l'argent, je, je le vois et je le mesure mais enfin les mots ont un sens. Les mots ont un sens, la trajectoire Ondam, notamment pour l'hôpital, elle est 2 fois plus ambitieuse et plus généreuse que ce qu'on a connu dans la décennie 2010 et certains sur ces bancs étaient présents, moi aussi, il se trouve que j'ai travaillé au ministère de la Santé à l'époque dans un précédent quinquennat ces moyens pour l'hôpital, on en aurait rêvé, on en aurait rêvé 4 virgule un % sur l'hôpital, c'est 2 fois plus qu'en moyenne sur la dernière décennie, et en plus on a une base plus importante puisqu'on allait 13 milliards d'euros du Ségur il y a pas une mesure d'économies sur l'hôpital, dans ce PLFSS pas une pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le budget de l'hôpital va dépasser les 100 milliards d'euros l'an prochain, on peut considérer qu'il faudrait que ce soit plus moi j'entends, mais parler d'austérité quand on a un budget de l'hôpital qui va dépasser les 100 milliards d'euros, quand on a un Ondam qui est d'oeuf qui va 2 fois plus vite que dans la décennie précédente, quand il y a pas de mesures d'économie qui, à 800 millions d'euros qui sont provisionnées au titre de l'inflation puisqu'évidemment, c'est une honnêtement ça ne me semble vraiment être en dehors de la réalité. Oui, les mots ont un sens, monsieur le Ministre, et quand les fédérations les toutes les fédérations hospitalières vous dit ce qu'il manque un milliard quand il manque un milliard ça veut dire qu'il faudra qu'elle fasse un milliard un milliard d'économies poursuivent l'évolution mécanique, on l'a déjà dit, du vieillissement de la population des pathologies chroniques de l'innovation médicale dans un contexte de forte inflation, notamment énergétiques mais pas qu'eux aussi qui touche le poste alimentaire s'il manque un milliard, s'il faut qu'elle fasse un milliard d'économies, cela s'appelle l'austérité, quel que soit le niveau dont dame que vous que vous présentez sur le plan facial. Allez je mais aux voix ces deux amendements identiques avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Rejeté. 5 amendements en discussion commune le 511 madame Meunier. Merci monsieur le Président, cet amendement propose une répartition de l'Ondam afin de prendre en charge en compte l'inflation et les besoins humains dans les secteurs sanitaire et médico-sociaux pour 2023, il permet notamment de financer la création des 15500 postes supplémentaires nécessaires en Ephad afin d'atteindre la trajectoire des 18500 préconisé notamment dans le rapport El Khomri pour des raisons de recevabilité le montant alloué aux objectifs de dépenses relatives aux établissements de santé est prélevé sur l'objectif des dépenses de soins de ville, laissant inchangé l'objectif des dépenses, cet amendement a été travaillé avec la FAP et l'une

Merci monsieur le président, il s'agit de 2 un budget pour la revalorisation des carrières des psychologues cliniciens en milieu hospitalier. Merci. Le six 89 madame Darcos défendu et bien sûr tout cela, madame la rapporteure faites au mieux. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ces différents amendements visent donc à modifier la répartition des dépenses entre les différents sous-objectifs de l'Ondam nos différents collègues veulent ici interpellé le gouvernement sur les niveaux des sous-objectifs avec des majorations proposée sur les sous- objectif relatif à l'hôpital ou au médico-social cependant l'état actuel de ce qu'est l'Ondam nouvelle ventilation des sous-objectifs n'aurait en réalité aucune portée normative sur l'affectation des crédits, l'avis est donc défavorable, modifier les sous-objectifs sans modifier la politique derrière ne conduirait qu'à affaiblir la sincérité de l'Ondam 2023, cela me permet une nouvelle fois utile de rappeler que la commission, comme elle l'avait souhaité l'engagé lors de la révision de la loi organique

monsieur le ministre, on ne peut approuver un objectif de 250 milliards d'euros avec 2 enveloppes de plus de 100 milliards qui ne sont pas plus précisément répartis c'est ce cela est sans commune proportion avec le budget d'État ou des programmes budgétaires sont parfois inférieur au milliard d'euros, et ce n'est plus viable, les parlementaires doivent être en mesure d'approuver une ventilation fine des dépenses cet enjeu démocratique, alors c'est un enjeu démocratique, alors que les recettes de l'assurance maladie, sont essentiellement des contributions et impôts, et que le pilotage des dépenses répond à des logiques de pilotage budgétaire qu'on le veuille ou non. Donc, avis défavorable sur sur l'ensemble, merci. Avis du gouvernement. Merci monsieur le président, on a évidemment tous à coeur de renforcer les moyens du secteur médico-social dans notre pays, qu'il s'agisse de la prise en charge des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap et c'est ce que prévoit ce Plfss avec 700 millions d'euros de plus par rapport à l'an dernier et puis je le dis avec un Ondam, encore une fois très ambitieux, très généreux 5 virgule 1 % sur les personnes âgées 5,2 % pour les personnes en situation de handicap, moi j'ai le souvenir, il y a quelques années 2015, 2016 c'était un pour 100 l'Ondam. Pour le médico-social pour les personnes âgées, un Là on est à 5 virgule 1 % c'est 5 fois plus, donc c'est extrêmement ambitieux et c'est extrêmement généreux, parce qu'on veut évidemment à accomplir les engagements de campagne qui ont été pris par le président de la République, son programme avec le recrutement de soignants dans les EPHAD avec les 2 heures de prise en charge de convivialité en plus pour les seniors à domicile avec des grands projets pour les personnes âgées, donc j'ajoute que ces amendements en plus rajoute des moyens sur l'Ondam médico-social mais en retire à due concurrence à l'Ondam sur la médecine de ville, alors je sais qu'il y a un enjeu de gage et évidemment de souhait de rester dans la même enveloppe mais très concrètement, ces 3 milliards de qui sont retirés à la médecine de ville, ça veut dire parce que on est pas dans des moyens financiers infini, on est dans une logique contrainte, moi je ne peux pas lever un gage à ce niveau-là, ça veut dire que si ces amendements ont été adoptés, a été définitivement adoptée à l'issue de la procédure, il faudrait des rembourser les consultations en ville pendant 2 mois pour faire l'économie correspondant aux 3 milliards de qui doivent être retirés à la médecine de ville, d'autant plus que vous avez dans des votes précédents supprimer des mesures d'économie pour la médecine de ville pour la ville, je pense notamment aux économies sur la biologie médicale qui ont été supprimés, il y a une taxe qui a été votée, mais ce n'est pas l'Ondam, oui, il y a une taxe qui a été votée en lieu et place, et ça n'est pas du coup l'Ondam, ce ne sont pas des économies sur l'Ondam une taxe supplémentaire et donc ça veut dire que l'effort sera encore plus important sur la ville, donc nous on est aussi attaché au secteur de la vie, la nos médecins libéraux consultations qui réalise qui doivent pouvoir continuer à être remboursé pleinement et toute l'année et donc pour toutes ces raisons, parce que l'Ondam médico-social est particulièrement ambitieux et par qui nous sommes pas justifiée de diminuer l'Ondam sur la ville, c'est un avis défavorable. Merci, nous avons d'abord Madame la rapporteure puis Monsieur Jomier comment non. Madame la rapporteure clôturera. Mais oui ah clôture. Merci monsieur le président Monsieur Nice, vous êtes venue rouvrir en fin de PLFSS une discussion de début du texte, alors désolé monsieur le président, mais il va falloir quand même falloir dire quelques mots d'abord vous avez reproché à mes collègues de vouloir supprimer un article qui est obligatoire au titre de la loi organique, vous avez raison, mais je vous rappelle que vous, le gouvernement a transmis au Sénat, un à un, PLFSS sans article 3 qui lui aussi obligatoire au type de la loi organique, et c'est le Sénat qui l'a rétablie dans une version qui ne nous satisfaisait pas mais qui au moins la rétablit donc ne donnez pas des leçons de respect de la loi organique aux parlementaires. Comme ça, c'est toujours risqué 2ème point c'est vous avez la mémoire des Ondam mais visiblement vous n'avez pas la mémoire de l'inflation depuis que les lois de finances de la Sécurité sociale existe depuis que l'Ondam existe jamais l'inflation n'avait été à ce niveau, on va terminer l'année entre 6 et 6 et demi % je ne sais pas exactement et en 2023 probablement autour de cinq alors voilà, vous vous venez répéter, répéter jusqu'à plus soif ah mais on avant, c'était un et demi de oui, mais l'inflation était jamais supérieures à deux voilà donc comparons ce qui est incomparable, tout ça n'a pas de sens, la vraie question, ce sont ces ce savoir si on répond et je souscris à ce que dit le ministre de la santé, la prévention là dessus : aux besoins de santé du pays par exemple pour ce qu'est la partie maladie et non pas mener une politique de l'offre, ça, c'est ça, c'est un débat qui est un débat intéressant et qui nous qui nécessite que nous changeons d'ailleurs le mode d'élaboration de la loi de finance de la Sécurité sociale et qu'on le fasse, précédé d'un débat sur les objectifs national de santé du pays voilà, remettons les choses d'aplomb et qu'en début de quinquennat vous arriviez avec un PLFSS aussi faible, aussi mal écrits, parfois un brouillon, mal cadré alors de d'au lieu d'arriver avec un texte qui, plus une nouvelle dynamique manque montre que votre quinquennat est déjà à bout de souffle. Merci. Bien, je vais mettre aux voix successivement les 5 amendements avec avis défavorable de la commission défavorable du gouvernement le 511 d'abord. Qui est pour.

le 800 81. Qui est pour, qui est contre. Le 689 qui est pour retirer, il a retiré. Madame la rapporteure, vous vouliez la parole sur l'article 47.

mes chers collègues, le vote de l'Ondam est un moment suffisamment important d'examen d'un PLFSS pour que l'on s'y arrête un instant, il s'agit d'approuver une prévision de dépenses de l'ordre de 250 milliards d'euros et rien de moins, certaines missions du budget de l'État, à elle seule donne lieu pour un 10ème de la somme à une discussion générale, or, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, rien de tel pour l'objectif national des dépenses d'assurance-maladie, la commission des affaires sociales du Sénat avait fait des propositions opérationnelles lors de la révision de la loi organique sur les lois de financement de la Sécurité sociale, l'an dernier, ces propositions avaient été balayé d'un revers de la main par le gouvernement et le rapporteur général de l'Assemblée nationale, on nous a opposé la facilité de gestion de la sécurité sociale permettant de donner en cours d'année, des milliards d'euros à Santé publique France et le fait qu'il n'était pas question de limiter le recours aux soins faute de crédits budgétaires, ce n'était pas du tout le sujet, mais vous aviez refusé de l'entendre, la commission avait aussi demandé une chose simple que ne soit plus une si grande enveloppe si tu peux préciser, nous discutons d'un Ondam de 250 milliards d'euros avec, nous l'avons déjà dit 2 enveloppes principale dépassant les 100 milliards d'euros, je le redis, n'est pas tenable de faire voter 100 milliards d'euros de dépenses sans que la ventilation de celle-ci ne puisse être précisée ni modifié par les parlementaires. Faute de telles évolutions, la Commission, par la voix de la présidente notamment et par les questions régulière que j'ai adressée à interroger le gouvernement sur plusieurs points d'une part, concernant les montants des arrondis à la centaine de millions d'euros ne sont pas acceptables, d'autre part, sur le fond, alors que de nombreux crédits de l'Ondam sont des enveloppes pilotable, c'est un enjeu démocratique que de pouvoir en connaître le montant avant le vote, or, alors que le pays est fortement préoccupé par la situation de l'hôpital, nous ne pouvons avoir de débat descend sur son financement, faute d'information, ainsi, alors que le financement de l'hôpital repose pour partie sur des dotations, pas de précision sur les enveloppes de dotation concernant les Miyake, pour les hôpitaux ni concernant les dotations populationnelles ou socle pour les hôpitaux de proximité ou encore les soins de psychiatrie, enfin, les investissements financés par la cadette ne sont ni dans le PLF ni dans le PLFSS enfin, Madame la Ministre, je voudrais partager avec vous et avec mes collègues, une interrogation : le ministre François Braun a annoncé il y a moins de 10 jours 400 millions d'euros de crédits supplémentaires sur les soins critiques et la pédiatrie une partie de ce montant, nous a conduit à réviser à la hausse l'Ondam 2022, mais le gouvernement nous indique, je cite, qu'il allait marges suffisantes pour absorber les mesures nouvelles en 2023, mais où sont ses marges, avait-on dans le texte, déposé un Ondam si confortable qu'il soit possible d'annoncer plusieurs centaines de millions d'euros de dépenses nouvelles, sans modifier les montants soient les annonces ne sont pas justes et il ne s'agit pas de rallonge soit l'Ondam, n'est pas correct, nous nous sommes lourdement interrogé en commission sur la crédibilité de l'Ondam 2023, force est de constater que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, que le gouvernement nous soumet aujourd'hui les 10 crédibles ni sincères pour ces raisons, la commission a adopté un avis à donner un avis défavorable à l'adoption de l'Ondam 2023 je vous remercie. Merci, je suis saisi. D'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains sur l'article 47. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Sur l'article 47 Votants 343 exprimés 323 pour l'article 24 contre l'Arctique 299 l'article 47 n'est pas adopté. Après l'article 47 le 115 ah, madame la présidente. je tenais à faire une imprécision bon Bernard Jomier là déjà évoqué, on nous dit en effet un rejet de l'Ondam, n'est pas possible parce que c'est un élément obligatoire de la loi de financement pour autant aucune disposition organique ne prévoit d'équivalence entre Roger l'Ondam et rejet du PLFSS par une assemblée en terme de procédure, l'article L L O 111 1 du code de la sécurité sociale n'impose que l'ordre d'examen des articles, des parties du PLFSS et que l'adoption de la 3ème partie avant l'examen de la quatrième, cette dernière disposition revient donc à considérer que le rejet de la 3ème partie, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs une fois et vaut un rejet de l'ensemble du PLFSS en reprenant la décision de 1979 le Conseil avait considéré que la nécessité d'adopter la première partie de la loi de finances avant de passer à l'examen de la 2ème partie ne faisait que tirer les conséquences au plan de la procédure législative du principe fondamental selon lequel il faut garantir qu'il ne sera pas porter atteinte lorsque l'examen des dépenses aux grandes lignes de l'équilibre défini telle qu'il a été arrêté par le Parlement, rien de tel n'existe pour les objectifs de dépenses et pour la dame qui figure en 4ème partie, on peut d'ailleurs établir une analogie avec le rejet de telle ou telle mission dans le cadre de la loi de finances, qui n'empêche pas l'adoption du texte, il semble donc bien au Sénat de mettre, on voit l'ensemble de la 4ème partie

Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Commission avait souhaité dans le cadre de la révision de la loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale inscrivent une série de clauses de retour devant le Parlement en cas d'écarts constatés en cours d'exercice par rapport aux trajectoires de recettes ou de dépenses voté aussi le présent amendement vise à préciser cette exigence dans le cas de l'Ondam 2023 un dépassement de l'Ordre de de 5 milliards d'euros conduirait le gouvernement à venir présenter à la commission des affaires une trajectoire sur laquelle elle serait chargée d'émettre un avis pour rappel, l'Ondam 2000 22 et réviser dans ce PLFSS pour plus de 9 milliards d'euros, sans que ces dépenses anticipées dès avril n'avait été présenté devant le Parlement. J'ai le président madame la rapporteure votre amendement est déjà satisfait donc un un retrait sinon avis défavorable dans son avis du 30 mai d'ailleurs, le comité d'alerte de l'Ondam a d'ailleurs fait état d'un risque sérieux de dépassement de l'Ondam 2022 supérieure à 0 5 et la notifié au parlement donc votre normalement moment comme je l'ai dit déjà satisfait en pratique et donc j'y suis défavorable. Moi ce que je voulais dire c'est qu'à chaque fois on nous dit ça, mais il y a le comité d'alerte et la Commission des comptes de la Sécurité sociale mais ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le Sénat, donc désolé, on le dit à chaque fois. C'est dit, c'est dit Monsieur Savary. Ben oui, mais moi c'est un putain de président de de de l'Mecque, ce que je souhaitais intervenir puisque Monsieur le Ministre. Vous avez donné un avis défavorable allez-y, allez-y Monsieur Savary c'est quand même une somme importante, me semble-t-il, hein, je voulais rappeler en quoi consistait la procédure, le gouvernement devrait adresser sans délai aux commissions des Affaires sociales et de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport qui présenterait les raisons de la dégradation de la situation financière de la sécurité sociale, les modifications projetées des tableaux d'équilibre Italie établi dans la pression de lois précédentes lois de financement et des objectifs de dépenses, ainsi que les mesures envisagées de redressement des comptes de la Sécurité sociale pour l'année en cours à partir de là, les commissions des Affaires sociales, Assemblée, Sénat ferait connaître leur avis au Premier Ministre sur les modifications et les mesures évoquées précédemment, monsieur le Ministre, pourriez-vous donc nous préciser à partir de quel moment de dépassement de l'Ondam vous estime rien tenu d'adresser un tel rapport au Parlement et ça à hauteur de 5 milliards de 10 de 20 de quarante ou bien considérez-vous que le vote des objectifs de dépenses en loi de financement de sécurité sociale et le nouveau cadre organique ne Servent à rien ou ne vous lie en rien plus globalement cet avis défavorable vient après d'autres avis défavorable à des amendements proposent proposant de fixer dans la loi les crédits des agences à tirer les conséquences en loi de financement de sécurité sociale des conventions médicales et même à vous donner des outils. De maîtrise des dépenses dont vous pourriez user ou non hier à votre guise, comme la possibilité de refuser une convention qui s'écarterait trop de l'équilibre, voté en loi de financement.

de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. 100 15 de la Commission avis défavorable du gouvernement oui qui est contre.

Merci Monsieur le Président, alors cet amendement demande un rapport, nous sommes en plein suspense en vue d'instaurer une loi de programmation pluri-annuel de l'Ondam et de reconnaître son caractère stratégique en effet le Ségur de la santé a conclu sur la nécessité de donner un cadre. Pluriannuel à l'Ondam, celui-ci existe déjà pour partie en ce qui concerne les ressources des établissements de santé à travers cet amendement s'expriment le besoin que la programmation pluriannuelle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, intègre les missions d'intérêt général, financé par le fonds d'intervention régional et accorde au Parlement une visibilité dans le domaine aussi médico-social, une véritable visibilité au-delà des insuffisante grandes lignes budgétaires du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 2027 dans lequel est indiqué pour seule perspective en matière de Ondam une progression générale à hauteur de 3 septembre 2023 de 7 en 2024 puis en 2025, sans plus d'informations quant quant aux évolutions à l'intérieur même de cet objectif global au delà de ce cadre général des financements dédiés à la recherche et à l'innovation ont depuis de nombreuses années, servi de variable d'ajustement à la régulation comptable de l'Ondam pour éviter de retomber dans une nouvelle phase d'érosion progressive des moyens fléché, ou du moins d'approfondissement de cette érosion alors des moyens fléché au financement de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, nous en appelons à prévoir l'évolution des crédits sur la durée en on la calant a minima sur le taux de l'évolution de l'Ondam hospitalier. Merci, avis de la commission. Ce sera un avis défavorable, monsieur le Président sur la psy on on fera un suivi ma chère collègue et sur les SSR, nous allons-y revenir avec un amendement du gouvernement. Merci, avis du gouvernement.

Avec 2 avis défavorable est pour. Qui est contre, rester. Le. à un amendement un sous-amendement l'amendement du gouvernement, Madame la Ministre, le 1100 Oui, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, tout d'abord, le gouvernement revient devant vous avec cet amendement concernant la réforme du financement du SSR, nous avons eu le débat jeudi j'avais déjà regretter que cet amendement de prolongation de la mise en place de la réforme puisse revenir devant vous, cet amendement est arrivé tardivement, je m'en suis excusée, mais ceci est un moment est arrivé tardivement de devant vous, c'est bien parce que nous essayons, avec tous les acteurs de pouvoir faire aboutir cette réforme dont, je le redis, nous y tenons et vous y tenez, nous y tenons tous simplement vraiment des difficultés techniques ne permettaient pas que cette réforme soit applicable partout et sur tout le territoire, au 1er janvier nous vous avions proposé un amendement de d'un report d'un an, nous revenons vers vous avec la volonté de pouvoir d'abord entendre ce que vous nous avez dit en disant que ça fait plusieurs fois qu'on reporte et qu'il ne fallait pas aller plus loin, néanmoins, j'insiste sur le fait que nous souhaitons d'abord petite hein, que cette réforme soit mise en place, je crois que c'est une volonté partagée mais nous souhaitons aussi qu'elle soit mise en place dans les meilleures conditions, partout sur le territoire en même temps ce pourquoi nous sommes arrivés très tardivement devant vous, c'est que nous essayons toujours de travailler avec les opérateurs, mais il est évident que nous ne pourrons pas la mettre en oeuvre partout et en même temps sur tout le territoire, je sais votre volonté d'égalité d'accès et nous vous proposons un nouvel amendement avec un report de de 6 mois pour la mise en place de cette réforme du SSR qui est nécessaire et nous le savons tous. Merci le sous-amendement 1145 madame la rapporteure.

vous l'aurez noté alors ce ce nouvel amendement pas si nouveau, mais nouveaux quand même puisqu'il vise à organiser ce qui pourrait ressembler à une seconde délibération dans notre hémicycle sur un sujet déjà traité à l'article 25, le gouvernement avait déposé mercredi un amendement de dernière minute visant à reporter une nouvelle fois l'entrée en vigueur de la réforme du financement des soins de suite et de réadaptation, cette réforme, qui devait intervenir en 2021 avait été reporté en loi de financement de la Sécurité sociale 2021 en raison de la pandémie reporté en 2022 elle avait à nouveau été reporté, je l'avais rappelé le jeudi lors du dernier PLFSS par le biais d'un amendement de dernière minute encore jeudi matin, le Sénat a rejeté la demande un 3ème report du gouvernement qui entendait à nouveau repoussé l'entrée en vigueur, cette fois en 2024 donc 2 raisons ont conduit à ce rejet est une raison de de méthode et et vous pouvez le comprendre peut pas chaque année demander cette semaine avant l'entrée en vigueur prévue un report d'un an, une autre de fond, nous avions estimé que le report successifs commençait à devenir le signe d'un enlisement, voire un abandon de la réforme qu'il n'est nullement souhaitable cette réforme est nécessaire et son entrée en vigueur rapide est indispensable, j'ai pu échanger à plusieurs reprises que la ministre et ministre de la Santé à ce sujet, la commission des affaires sociales du Sénat n'est pas aveugle aux difficultés éventuelles des établissements ou aux difficultés techniques techniques des agences régionales de santé qui sont durement mobilisés par une pandémie qui dure, le gouvernement nous propose aujourd'hui un report de 6 mois de la réforme, dont acte, j'estime qu'un report de cette heure d'être acceptable au regard des discussions que nous avons pu avoir, je considère qu'il est acceptable aussi pour 2 raisons, par esprit de responsabilité, d'une part mais aussi d'autre part parce que ce délai ne correspond pas à l'examen du prochain Plfss donc comme ça on aura pas un amendement de dernière minute, l'année prochaine en novembre 2023 cependant, si cet amendement est acceptable, il est à certaines conditions et je souhaite que le gouvernement s'engage tout d'abord à tenir cette ligne à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire clairement à de ne pas modifier cette échéance, à l'occasion de l'utilisation d'un nouveau 49 3 à tenir l'échéance d'autre part, en prenant les mesures réglementaires nécessaires dès le début de l'année et en garantissant d'un point de vue opérationnel, l'entrée en vigueur au 1er juillet au plus tard,

un amendement visant à ajuster la rédaction en précisant que la date au plus tard le 30 juin 2023 je formule une dernière observation quant à cette entrée en vigueur concernant la transition, nous avons été alertés sur les évolutions des ressources simuler que certaines régions considérées insuffisantes pour le maintien de l'offre de soins, c'est le cas notamment des établissements d'Île-de-France avec ce report sur report Madame la Ministre, le gouvernement n'a pas mené à bien la transition qui était prévu, n'a pas prévu de lissage progressif, vous comptez faire entrer la réforme d'un coup, sans transition, or les précédents je pense là à la réforme tarifaire des Ephad il y a quelques années, nous invite à la prudence, vous l'aurez compris madame la Ministre, cette réforme est souhaitable et souhaitée par le Sénat. Et donc c'est un avis favorable à votre amendement sous-amendé par l'amendement de la commission. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement sur le sous-amendement. Donc un avis favorable au sous-amendement et je remercie la responsabilité de la commission des affaires sociales pour l'entrée en vigueur, et pour nous accompagner sur l'entrée en vigueur effective de cette réforme nécessaire, dont nous savons tous qu'elle est nécessaire. Hé bien. Donc nous avons un sous-amendement oui madame. Oui, bon, j'étais intervenu moi oui effectivement pour la suppression du report tout simplement en faisant là pour le coup, l'écho de la Fédération hospitalière de France et de la FEHAP,

non lucratif par rapport au secteur privé lucratif de mode de financement différent, c'était, vous l'avez dit, un enjeu d'équité, enfin ou d'égalité là peut le mot et plus juste qu'il fallait reprendre en compte et puis il y avait des avancées, comme la prise en compte de la dotation populationnelles tout ça sur lesquelles par

qu'on avait effectivement parlé d'une crainte d'un nouveau report, voire d'une écoute, un peu plus, je me souviens de ce que j'avais dit, plus attentive à la volonté de la fédération privé lucratif de, de, d'avoir un nouveau délai, on avait peur d'une décision donc et moi je me réjouis, hein, de, de, d'un report, simplement si un si moi, effectivement, comme l'a pointé Madame la rapporteure parce que on exclut de ce fait un nouveau report lors d'un prochain Plfss alors personnellement, enfin le groupe écologiste votera ces amendements. Bien. Allez, je vous envoie le sous-amendement et l'amendement donc en accord, le gouvernement et Commission sous-amendement d'abord le 1145 et pour. Merci, amendement 1144 sous-amendé ainsi. Qui est pour, qui est contre, ils sont donc adopté. à l'article 47 bis Madame Imbert, l'amendement 116. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, pour la 3ème année consécutive, le gouvernement prévoit que le comité d'alerte n'aurait plus à alerter en cas de dépassement du montant voté cette année dans le cas où le dépassement résulte de la crise, force est de constater qu'alors que les dépenses d'assurance maladie, subissent les effets de la pandémie, puis du contexte inflationniste, le rôle d'alerte n'est plus d'actualité, cependant, alors que la commission regrette à nouveau la faiblesse des données disponible sur l'exécution de l'Ondam, en cours d'exercice, la mission d'information du comité est nécessaire aussi, alors que le pilotage gendarmes ne semble plus d'actualité pour le gouvernement, il est proposé de changer la dénomination du comité d'alerte en comité de suivi de l'Ondam. Madame la rapporteure vient de faire la réponse défavorable car oui, contrairement à ce que votre amendement laisse supposer le rôle d'alerte du comité n'est absolument pas suspendu par l'article 47 bis de ce PLFSS le comité devra bien continuer à notifier, notamment au Parlement tout risque sérieux de dépassement d'ampleur de l'Ondam si on dames, il y a d'ailleurs et d'ailleurs, il a fait le 30 mai 2022 en alertant le Parlement sur le risque de dépassement de l'Ondam. Merci. Je mets aux voix donc le 100 cesse de la Commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient, il est adopté, je mets aux voix, l'article 47 bis qui est pour. Qui est contre. Il est adopté à l'article 48 je suis saisi d'une demande de parole Madame Jasmin. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, ma prise de parole concerne le plan chlordécone l'action du gouvernement va dans le mon sens et l'Opecst l'a confirmé récemment lors d'un bilan d'étape, il est indispensable aujourd'hui que vous puissiez accompagner les familles accompagner de la communication pour que la bonne ces formations circulent accompagnés également avec l'aide de la Caisse Générale de Sécurité sociale, pour que les les familles et particulièrement les femmes et la possibilité de remplir les documents pour les enfants également, il est nécessaire pour, surtout pour ceux qui sont dans des situations avec des situations difficiles, avec des problèmes endocriniens, que vous connaissez, il est aussi important qu'il y ait un accompagnement, il faut également impliqué les associations toutes les associations qui, depuis, tantôt se sont élevées, mais qui sont aujourd'hui très volontaire pour le nous l'avons vu avec l'Opecst, une association de la Martinique et une de la Guadeloupe ont été auditionnés, nous les avons entendus, donc ça va dans le bon sens mais il ne faut pas faire de n'importe quelle manière il faut vraiment les acteurs et prendre les mesures pédagogiques nécessaires pour que l'adhésion de l'ensemble de la population de nos territoires, Guadeloupe et Martinique soit réelle, je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président, les dotations afférente au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comme celle d'ailleurs alloués au Fonds de cessation dissipés de l'activité des travailleurs de l'amiante très sensiblement constante d'un PV à l'autre, se pose toujours la question de la reconnaissance des expositions et du procès de l'amiante, mais le débat ne pose, ne se pose pas ici ma collègue Katia pour ce pôle, il a d'ailleurs déjà eu l'occasion d'écrire au garde des Sceaux à ce propos, les membres du groupe CRCE comme beaucoup d'autres, n'oublie pas les victimes de l'amiante, mais je voudrais saisir ici l'occasion de cet article pourrait Vicky pour éviter un autre scandale l'empoisonnement au plomb par les industries qui perdure dans le temps, nous avions déposé 3 amendements à ce sujet pour faire reconnaître le saturnisme comme maladie professionnelle, y compris pour les riverains exposés sans avoir été nécessairement salariés l'indemnisation de cette reconnaissance, et enfin la prise en charge complète dans le cadre de parcours de soins avec des spécialistes sans dépassement d'honoraires, hélas, ces trois amendements été déclarée irrecevable et cette prise de parole veut attirer l'attention du gouvernement, Madame la Ministre, sur ce drame pour prendre un exemple, cher à ma collègue, Katia pour il y a de nombreux enfants qui sont atteints de nombreux enfants qui sont atteints de saturnisme de l'eau dans le Pas-de-Calais et d'ailleurs pas que des enfants, il y a également des adultes et des jeunes qui ont un taux de plomb qui est bien supérieur donc nous pensons au niveau de, de, du groupe CRCE, qu'il faut vite prendre des mesures d'état en quelque sorte, qui passe par l'assainissement des sols mais également par l'indemnisation de ces personnes et de leurs familles et en tout cas, cette prise de parole et l'occasion, madame la ministre d'attirer une fois de plus plus votre attention sur ce drame. Oui, merci, monsieur le Président, Madame la Ministre, alors cet amendement, moi je dirais c'est un amendement habituel annuelle, voilà, oui c'est ça, vise à diminuer de d'ici, de 200 millions d'euros, le transfert de la branche AT-MP accidents du travail-maladies professionnelles à la branche maladie au titre de la sous-déclaration

et ce montant constitue le bas de la fourchette proposée par le dernier rapport de la commission chargée d'estimer tous les 3 ans, le coût pour l'assurance maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais cette estimation, elle reste quand même sur une base statistique, or pour une large part, ce phénomène de sous-déclaration résulte de décisions et de comportement qui échappe à la branche AT-MP ses principaux facteurs sont l'insuffisance de la formation des médecins, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, la mauvaise information des patients, la complexité des procédures ou encore les contacts trop peu développée entre la médecine de ville et la médecine du travail, ce transfert, c'est un très mauvais message envoyé aux entreprises qui ont fait des progrès importants en matière de risques professionnel comme le montre la diminution par exemple de 10 pour 100 des maladies professionnelles entre 2012 et 2021 et par ailleurs tout se passe comme si la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention santé au travail n'a apporté aucune amélioration, je demande aussi à voir les statistiques sur ce qu'on pourrait appeler la sur déclaration ou sur Reconnaissance des AT-MP qui n'est pas établie alors dans ce contexte, l'augmentation de ce versement apparaît comme une ponction réalisée dans des conditions peu transparente et comme une contribution visant à combler une partie du déficit de la branche maladie, j'aurais 2 questions est-ce que vous pouvez imaginer qu'une autre caisse soient tenus de payer le coût supposé du non-recours aux prestations qu'elle est chargée de verser et enfin ce que nous préférions ce serait de flécher ces montants sur la prévention et l'accompagnement des patients, salariés des médecins ou de maladies comme vient d'en d'en parler Madame Cohen. Merci madame la ministre. Monsieur le président, madame la rapporteure, vous l'avez dit, le gouvernement a fait le choix d'atteindre progressivement la borne basse de l'estimation dans le respect de la démarche scientifique scientifique, je le précise, et de l'équilibre de la branche, une première étape a eu lieu dans la FSS pour pour 2022, qui a porté ce transfert à 1 virgule 1 Myriam le montant pour 2023 de virgule 2 milliards s'inscrit dans la continuité de ses démarches qui avait déjà d'ailleurs été annoncé au sein de la FSS 2022, à cet égard une réduction du montant de transfert ne paraît pas opportune elle reposerait sur aucun fondement scientifique et irait à l'encontre des études disponibles, nous sommes donc défavorable à votre amendement pour répondre sur la chlordécone, vous le savez, madame la sénatrice, nous nous sommes réunis la semaine dernière, puisque le le le ministre Jean-François Carenco et et moi-même suivons de très près le développement du plan corps déconne et à cet égard le Conseil le grand conseil scientifique qui aura lieu du 12 au 14 décembre marquera une part importante et notre volonté de communiquer de façon très pédagogique à la à l'égard de nos concitoyens aux Antilles est importante et donc nous savons qu'il faut aller encore plus vite et accompagner les habitants des Antilles sur ce sujet et nous partageons avec vous, le développement de ce plan chlordécone si important. Merci madame pour mange.

on parle d'un d'une estimation basse, comme l'a rappelé : Madame le Ministre, d'arrêt de travail qui ont été déclarées à l'assurance-maladie, comme des un arrêt de travail maladie ordinaire, je serais tenté de dire. Et dont on estime, par une évaluation basse toujours qu'ils auraient dû faire l'objet d'un arrêt de travail. Du soit un accident de travail soit effectivement à une maladie professionnelle non non reconnue, dans un tableau, mais pas pas évaluer donc ça fait bien partie de la soul Reconnaissance des AT-MP dans laquelle sous-reconnaissance une partie et la sous-déclaration d'arrêt qui de fait donc son son des arrêts dont la charge a été porté par l'assurance maladie alors qu'ils auraient dû être portés par la TMP donc moi moi personnellement ce que je vois comme problème, c'est que là-dedans, c'est les salariés qui ont eu des arrêts maladie, simple, qui sont vraiment pénalisés parce que si la TMP les avait pris, elle paye là les 3 jours de carence elle majore les indemnités, il y a une meilleure invalidité,

moi je ne suis pas choqué par ce transfert, je suis la seule mais j'assume, et toujours est-il, si il y a des moyens à mettre, c'est pour qu'on mette fin à cette distorsion qui fait qu'un certain nombre d'arrêts de travail maladie sont de fait plutôt des des arrêts de travail qui aurait dû être traité en AT-MP. Allez, madame la présidente Gruny. Moi, j'entends bien ce que dit ma collègue et effectivement les les salariés n'ont pas été pris en charge correctement, donc moi ce transfert, c'est aussi un appel pour dire que cet argent doit rester dans la branche pour justement améliorer l'accompagnement des médecins, l'accompagnement des salariés mais, là, de faire le transfert, ça change rien parce que c'est même pas fléché juste justement sur de la prévention, mais sincèrement c'est pas ne pas payer, c'est c'est plutôt payer correctement et puis aussi parce que compte quand on l'entreprise ne connaît pas justement le le la maladie professionnelle, ben elle ne met pas en place non plus les dispositifs pour qu'il y ait pas d'autres salariés qui soit malade, donc voilà, moi je, je trouve que ce transfert c'est facile parce que finalement s'attaque pas à la cause. Bien, merci, allez je mais aux voix le 117 de la Commission, avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté, je mais aux voix, l'article 48 qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Après l'article 48 2 amendements identiques Madame Cohen le 771. Oui, monsieur le président, en France, une personne sur 5 est chaque année touché par un trouble psychologique, psychique, soit 13 millions d'individus des entreprises donc doivent prendre en compte effectivement ce nouvel enjeu de santé publique qui s'est d'ailleurs exacerbée avec la crise de la Covid d'autant plus que les chiffre sur le sujet sont préoccupants ainsi 34 % des salariés se sentent en situation d'épuisement professionnel, l'épuisement se traduit par différentes formes, une importante fatigue physique et émotionnel des troupes de l'humeur des troupes de la tension, une perte de motivation, voire d'enthousiasme au travail, selon un sondage récent 90 pour 100 des Français estiment que leur travail peut impacter leur santé mentale cette situation en progression constante, n'entraîne pas de réaction à la hauteur des enjeux ni de la part du gouvernement, ni de la part des entreprises cet amendement reprend donc une recommandation du du rapport d'information parlementaire sur l'épuisement professionnel qui date de 2017 afin que la commission chargée d'apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liés au travail actuellement supportés par l'assurance maladie, je vous remercie. Merci madame Jasmin le 1086 défendu merci. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, alors la commission qui est gentil, chargée d'évaluer le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des AT-MP a réaliser dans son dernier rapport rendu en 2021 une première estimation du coût de la sous- déclaration des pathologies psychiques toutefois la considérer que cette évaluation présentée encore des fragilités méthodologique hein liées au caractère multifactoriel de ces pathologies et n'a pas formellement intégré secoue dans son évaluation du coût global de la sous-déclaration, elle a d'ailleurs situés secoue dans une fourchette très très large comprise entre 73 et 287 millions d'euros, alors il est pas utile d'inscrire dans la loi un type de pathologie qui est déjà pris en compte par la Commission sous-déclaration, il est de surcroît prématuré de lui imposer de l'intégrer dans son évaluation globale

Merci madame Cohen j'ai bien entendu, donc on va retirer notre notre amendement mais on voit bien que la la fourchette qui est donnée par cette dernière étude est telle tellement large que ça nécessite quand même un soutien au niveau du gouvernement pour affiner les choses et de donner des les moyens suffisants, donc on le retire par rapport à ses explications, mais on voit bien qu'on a soulevé un problème réel et que ça nécessite une intervention beaucoup plus forte, je vais dire mais j'ai entendu au travers des propos de la ministre qu'elle comptait s'y atteler, donc je vais à en fin de ce de cet examen prendre ça comme un avis positif et retirer mon amendement. Madame Jasmin, vous le maintenez-vous retirer. Thierry également merci. Je mise aux voix, l'article 49 qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Après l'article 49 951 madame Poncet mange. Oui, je maîtrise pas bien la différence qui fait que ce soit par mais bon ça fait quand même reprendre ce cet amendement alors décrit comme un syndrome résultant d'un d'un stress chronique au travail, l'épuisement professionnel est un processus de dégradation du rapport subjectif de l'individu à son activité, je me permets, Madame la Ministre, une petite incise cette pathologie ne donne pas nécessairement en cas d'arrêt. Travail une prescription de médicaments ou d'actes de kiné, hein, par rapport aux arrêts sans prescription, donc vous avez tout à l'heure, dénoncer le l'augmentation par la télé consultation. Donc, je reprends depuis le 1er janvier 2022 il est intégré par l'OMS dans la nouvelle classification internationale des maladies comme un phénomène lié au travail en France selon les chiffres d'une enquête menée par opinion Way en 2021 2 5 millions de salariés seraient actuellement touchés par un syndrome de burn-out et de salariés sur 10 seraient en arrêt maladie pour des raisons psychologiques ayant trait à la fatigue professionnelle. Ce chiffre en constante augmentation sont en concordance avec l'imposition de plus en plus intenses, de nouvelles pratiques de management dans les entreprises qui usent, mais abusent souvent de l'engagement psychique. Et physique de leurs salariés, la perte de solidarité entre les salariés liés à la fragilisation des collectifs de travail et l'augmentation de la charge de travail, le stress aussi que du du temps mine la santé mentale de nombreux travailleurs sous le coup d'injonctions quelquefois paradoxal pourtant l'épuisement professionnel n'est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle, un phénomène lié au travail touchant autant de travailleurs doit pouvoir être reconnu par les pouvoirs publics afin d'être dûment pris en charge et que les salariés ne soient plus seul face à ce mal en progression, alors je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas explosé en même temps que mes, mes collègues. Oui. Allez, avis de la commission.

le nombre de maladies psychiques reconnues comme maladie professionnelle et c'est vrai en augmentation continue depuis 10 ans, la loi prévoit en effet explicitement que ces pathologies peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, via le système complémentaire. De reconnaissance hors tableau, en revanche, les troubles psychiques sont des pathologies pluri-factorielles dont il ne paraît pas possible de présumer qu'elles ont une origine professionnelle à partir de critères prédéterminés c'est pour ça que c'est difficile de les intégrer dans un tableau, c'est-à-dire on n'est pas contre, mais on préfère laisser ça aux commissions ils qui vont faire le le en plus l'augmentation de l'épuisement professionnel, moi je préfère, je préfère parler de ça, mais vous savez les liée aussi à l'épuisement général qu'on voit aussi chez les personnes en dehors, en dehors du travail et qui ont pris beaucoup d'ampleur aussi avec le confinement, donc, on retrouve aussi ça bien entendu dans dans l'entreprise, donc c'est un avis défavorable. Merci. Le gouvernement. Monsieur le président, madame la rapporteure, madame la sénatrice le gouvernement attache une très grande importance à la prévention et la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies. Psychique de plus, plusieurs années d'ailleurs, de nombreuses actions ont été menées par les pouvoirs publics en lien avec les partenaires sociaux dans le cadre du conseil d'orientation des conditions de travail pour faciliter leur reconnaissance dans le cadre de la voie complémentaire des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, d'ailleurs, leur nombre est en augmentation depuis plusieurs années puisque 1635 ont été reconnus en 2021 contre 1077 en 2019 les données en 2019 les données scientifiques actuelles ne permettent pas d'envisager la création d'un tableau qui instituerait une présomption d'imputabilité au travail dans ces conditions, le gouvernement est défavorable à votre amendement. Merci. Je mais voit le 951 avec 2 avis défavorable qui est pour.

qui revient sur le cumul emploi-retraite, qui permet aux retraités du régime général de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de secte à qui dites et avec ces pensions de retraite, le cumul peut être totale ou partielle, selon la situation du retraité, mais dans le cadre du cumul partiel emploi-retraite il faut attendre 6 mois pour reprendre une activité salariée chez son dernier employeur alors qu'il est possible de reprendre immédiatement une activité chez un autre employeur ça peut être et pour exactement la même fonction, mais pour qu'il y ait pas d'effet d'aubaine, cet amendement propose de supprimer ce délai de 6 mois pour permettre aux salariés proches de la retraite de garder leur emploi à condition qu'il soit à temps très partiel tout en diminuant progressivement, donc leur temps de travail, c'est une façon finalement de d'aller vers une retraite progressive qui est recommandé. oui, de la commission, monsieur le rapporteur. écoutez c'est c'est effectivement quelque chose d'intéressant qui mérite d'être étudiée dans le cas de la réforme des retraites, c'est la raison pour laquelle nous avons donné un avis défavorable et un certain nombre de propositions effectivement à faire à faire parce que ce sont des situations à envisager, il ne faut pas non plus qu'il y a un effet d'aubaine, hein, parce que sinon on pourrait penser qu'un employeur disent régulièrement allez vous mettez à la retraite et puis je vous bon donc à analyser mais à. Voilà. Alors c'est à vie quoi défavorable, très bien habillé du gouvernement. Les débats devront s'ouvrir dans le cadre des négociations menées par mon collègue Olivier Dussopt sur la réforme des retraites, donc un avis défavorable. Il est retiré, merci monsieur Fiole air et le cent

Donc défavorable, défavorable, très bien, alors je mets aux voix le 118 de la Commission, avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

se dérouleront le mardi 15 novembre à 14 heures 30, je vous rappelle également que je suis saisi d'une demande de scrutin public sur la. 4ème partie donc le vote va avoir lieu immédiatement, il y a des demandes oui, alors allez-y monsieur lévrier. Merci beaucoup pour une rapide explication de vote j'avais apprécié au début de ce Plfss le la volonté de professionnalisme de mes collègues qui ont réintégré les 2 premières parties de du PLFSS j'ai été particulièrement surpris de la fin de ce Plfss sur l'Ondam en particulier puisqu'en moins de 3 minutes en moins de 2 minutes, la commission et l'Assemblée ici à voter de contre, de suppression de l'article 47 proposée par Madame Cohen-puis par Madame Poncet mange et quelques minutes après, nous avons soi-disant au nom de la commission là que la commission ne votent que des amendements et pas des articles voter contre la même PLFSS dont vous avez voté contre et pour, en moins de 3 minutes, plus de 240 milliards d'euros, ce qui fait que nous abstiendrons sur cette 4ème partie. Madame la rapporteure générale. Oui, monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je voudrais, moi en tout tout d'abord remercier la qualité du travail mené ici au Sénat sur l'ensemble des des il y a eu des propositions des points de vue différents mais le le le débat s'est toujours passé de façon très très constructive, on s'est écouté on sait respecter, alors c'est vrai que moi je regrette toujours que finalement on discute d'un budget qui est 5 fois celui du de la défense en une semaine alors qu'après on va passer 2 semaines sur le budget, le PLF mais en tout cas je voudrais d'abord saluer le travail qui a été fait sur tous les bancs, je voudrais aussi remercier les ministres qui se sont succédé au banc, ils ont été toujours très, très présent, parfois ils étaient, ils étaient même deux et je dois dire qu'ils ont apporté des réponses sur un certain nombre de questions que nous leur avons posé je, je trouve que vraiment c'est à saluer je voudrais aussi remercier leurs collaborateurs qui nous ont également répondu pendant l'ensemble de cet examen, alors je me tourne maintenant vers l'ensemble de mes co- rapporteur, si je puis dire, pour leur leur dire combien j'ai apprécié de travailler avec eux, je voudrais également remercier la présidente de la commission des affaires sociales, l'ensemble des administrateurs autour de Delphine Mancel qui ont évidemment travailler toujours avec beaucoup de de célérité, on était quand même dans un agenda très très fermé et c'est vrai qu'il a fallu vraiment s'investir pleinement en très peu de temps, donc merci à vous toutes, à vous tous et puis rendez-vous Merci, j'ai donc été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains sur la 4ème partie du PLFSS il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56, le scrutin est ouvert.

le scrutin est clos. Parti votants 343 exprimés 305 pour 213 contre 92 la 4ème partie du PLFSS et adopté, mes chers collègues, je vais lever la séance, la prochaine séance est prévue le lundi 14 novembre à 18 heures pour le débat sur l'enseignement professionnel,

extrêmement nombreux, mais nous étions quand même là et remercier l'ensemble des rapporteurs pour. L'examen de ce texte, je vous remercie bien sûr la l'équipe de la Commission et les administrateurs c'est un PLFSS toujours un temps très contraint, cette année, ça l'a été encore plus je pense que nous avons eu néanmoins des débats apaisés, même si, même si. Martin lévrier nous dit qu'on n'est pas très professionnel, mais néanmoins, nous avons des bons débats apaisés, je remercie l'ensemble des. Des ministres qui se sont succédé au banc et Agnès Firmin Le Bodo ici présente et remercie la séance merci et à samedi non alors ce mardi. à mardi à mardi allez rien, madame la présidente, il est temps de rentrer la séance est levée.